monsieur le président.

C'est autant de moins pour la construction, la réhabilitation, les démolitions, le désamiantage dans nos territoires. Or il y a là un effort particulier à faire.

aux redéploiements internes pour trouver un meilleur équilibre.

d'une mise en attente de l'avenir de la participation de l'État au financement du régime de solidarité de Polynésie française, pour 12 millions d'euros, et de la fin du financement du projet de restructuration du service oncologie de Papeete. Si je comprends

mais, chaque année, il est insuffisant et ne reflète pas la réalité des risques. Comme l'avait souligné le rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur les risques naturels majeurs, il faut donner à ce fonds des moyens suffisants pour assumer sa mission de soutien d'urgence. Je propose donc de doubler les crédits qui lui sont alloués, afin de faire face aux aléas climatiques, qui sont de plus en plus fréquents. La

Le Fonds de secours a été fortement réévalué depuis 2015. En effet, la dotation allouée en PLF les années antérieures s'élevait à 1,6 million d'euros

en ressort que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses que dans l'Hexagone. Cet amendement vise à créer un fonds spécifique aux territoires ultramarins pour lutter contre ces violences. Il serait Il serait doté de 5 millions d'euros et aurait pour vocation d'accompagner les femmes victimes en les aidant dans la poursuite de leurs activités scolaires, professionnelles, en leur assurant un logement et une aide pour leurs démarches administratives. Le pilotage de ce fonds pourrait être confié aux associations qui collaborent déjà avec les préfectures. Quel est l'avis de la

Le Premier ministre a lancé le Grenelle des violences conjugales le 3 septembre. La semaine dernière

Laufoaulu, est retenu à Wallis en raison de la session de l'assemblée territoriale, vise à rappeler l'État à ses obligations issues de la loi du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer Des sommes considérables sont allouées dans le programme 123, sous forme de dotations spéciales, pour l'équipement scolaire en Guyane, et pour la construction et l'équipement des établissements scolaires en Guyane et à Mayotte.

est dans un état de délabrement indicible. Voilà quelque temps, un plafond s'est même écroulé dans une classe, mais heureusement en dehors des heures d'enseignement, ce qui a évité de déplorer des morts et des blessés. L'équipement scolaire est également très insuffisant : ainsi, les classes techniques ou professionnelles ne peuvent être assurées correctement, faute de matériel. C'est d'autant plus inadmissible que l'État a la charge financière de l'éducation, tant dans son fonctionnement que dans l'équipement et le bâti, à Wallis-et-Futuna. Cet amendement vise donc à faire face à l'urgence de rénovation du bâti scolaire et du manque d'équipements dans ce territoire en tendant à prélever 4 millions d'euros

Cet amendement vise à augmenter les crédits finançant le bâti scolaire à Wallis-et-Futuna. Son adoption entraînerait toutefois une baisse de l'action n° 04 du programme 138, créée dans le cadre du PLF pour 2019, et qui soutient des dispositifs grâce aux ressources dégagées par les réformes fiscales. Ces mesures spécifiques de soutien aux entreprises et associations ultramarines ont pour objet d'accompagner le développement économique et l'attractivité des territoires ultramarins. Les dispositifs ainsi financés concernent le prêt de développement outre-mer- élargissement des bénéficiaires et des critères d'attribution -, les subventions d'investissement dans le cadre d'appels à projets outre-mer, et le soutien au microcrédit outre-mer. Compte tenu de l'importance de ces actions, la commission des finances émet un avis défavorable.

puisque nous ne pouvons pas sortir de cette

On voit là, grandeur nature, les limites de l'exercice, avec cette façon de nous traiter dans un tiré à part. C'est un peu une tradition. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je ne partageais pas cet héritage, cette façon de faire. On a besoin d'une vraie révolution au fond.

n'est pas prise en charge, le dispositif n'est pas opérant, dans la mesure où les vols entre Nouméa et Paris sont tellement chers que les familles ne peuvent pas payer le complément. travers de cet amendement, que les plafonds soient revus pour être en cohérence avec le coût de la vie dans le territoire. Quel Je comprends les motivations des auteurs de cet amendement. Il est nécessaire de prendre en compte la situation des archipels et l'enclavement interne de certains territoires ultramarins.

En effet, les liaisons entre les îles de l'archipel néo-calédonien ne sont pas prises en compte en matière de continuité territoriale, alors que les liaisons entre les îles de Wallis et Futuna sont subventionnées au titre de l'aide à la continuité territoriale. La situation doit être la même pour nos collègues polynésiens. Il serait urgent de pouvoir agir sur ce point. De plus, le principe de continuité territoriale doit pouvoir s'appliquer pour les liaisons entre les îles d'un même bassin géographique, de manière à favoriser les échanges économiques.

Aussi, cet amendement vise d'abord à agir à la source, en créant un fonds spécifique, à hauteur de 500 000 euros, euros, afin de mettre à disposition des jeunes des moyens humains, matériels et financiers supplémentaires dans les établissements scolaires surchargés et de mettre en place un accompagnement périscolaire assuré par les adultes relais. relais. Concernant les adultes, ce fonds serait également dédié au financement des heures de formation centrées sur le cap lire-écrire-compter du compte personnel de formation (CPF) ou du conseil en évolution professionnelle auquel tout salarié a droit. Le pilotage de ce fonds pourrait être confié aux associations qui collaborent déjà avec les services des académies et Pôle emploi.

Madame la ministre, vous avez fait un effort, puisque vous avez élargi l'aide à la mobilité étudiante aux trajets effectués au sein d'un bassin géographique.

Je demande donc un transfert de crédits tendant à permettre la prise en charge intégrale des billets d'avion des étudiants qui ne sont pas boursiers pour les déplacements

Je comprends les motivations des auteurs de ces amendements. Il est peut-être nécessaire de prendre en compte la situation des étudiants qui paraissent trop riches pour être boursiers.

d'un quart des crédits destinés au financement des dépenses de fonctionnement du cabinet de Mme la ministre, de la direction générale des outre-mer (DGOM) et de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, ce qui paraît peu réaliste. L'avis de

(Ifrécor) joue un rôle important pour la préservation de nos récifs, qui sont menacés par le réchauffement climatique. L'année 2020 sera une étape charnière : pour le vingtième anniversaire de sa création, l'Ifrécor doit préparer son cinquième programme d'action. Elle doit réaliser un bilan de l'état de santé des récifs et des écosystèmes associés. Elle devra aussi répondre à l'objectif ambitieux de protéger 100 % des récifs coralliens français en 2025. Toutefois, les comités locaux font part d'un manque de moyens humains et financiers. je propose d'augmenter de 300 000 euros les crédits alloués à cet organisme. Il s'agit d'un effort modeste, mais nécessaire.

La part du fret dans les coûts d'approche est évaluée à 8 % si l'on considère le seul transport maritime, et à environ 15 % si l'on prend en compte les autres frais, dont ceux de manutention. L'aide au fret permet donc de diminuer le coût des importations. En outre, réformée par l'article 24 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, elle permet de développer le commerce inter-DOM. Cet amendement vise à accroître les crédits permettant l'insertion économique des départements et des collectivités d'outre-mer dans leur environnement immédiat. Pour ce faire, nous proposons d'augmenter l'aide au fret pour les produits importés des pays tiers et des départements et collectivités ultramarines,

Le présent amendement vise à augmenter le montant de l'aide au fret. Cette aide spécifique aux entreprises situées en Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles de Wallis et Futuna, permet de favoriser le développement économique ultramarin, d'améliorer la compétitivité dans ces territoires et de faire baisser les prix à la consommation.

Mme la ministre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2020, le montant des crédits de la mission « Culture » devraient s'élever à 2,96 milliards d'euros en en crédits de paiement. Cette somme ne reflète pas la totalité des crédits budgétaires affectés à la culture au sein du projet de loi de finances. Il convient en outre d'intégrer le montant de la dépense fiscale consacrée à la culture au travers de divers crédits d'impôt,

de 972 millions d'euros en crédits de paiement pour 2020. L'examen de ces crédits fait apparaître une diminution de l'ordre de 5 % des subventions accordées aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés en vue de la restauration des monuments historiques. Les crédits de Les crédits de paiement sont ainsi minorés de 7 millions d'euros entre la loi de finances pour 2019 et le présent projet de loi de finances. viennent financer le fonds incitatif et partenarial pour les monuments historiques des collectivités à faibles ressources, 2 millions d'euros vont, en revanche, alimenter le plan de mise en sécurité des cathédrales, lancé à la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je rappelle que les cathédrales sont des monuments historiques appartenant à l'État. Aussi, un risque pesant sur l'État se trouve financé par des crédits destinés à d'autres monuments qui ne lui appartiennent pas. Une telle option traduit un réel manque d'ambition. Cela étant, ce manque d'ambition s'inscrit dans le prolongement de la position adoptée par le Gouvernement concernant la cathédrale Notre-Dame de Paris, puisque ce plan ne donnera pas lieu à un geste budgétaire spécifique. Si la reconstruction de l'édifice est intégralement financée par le don privé, la sécurisation des cathédrales passera, quant à elle, par les collectivités territoriales et les propriétaires privés. S'agissant de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je m'interroge sur l'éventuelle réaffectation des fonds avancés pour les travaux de sécurisation, de déblaiement des gravois et d'enlèvement des échafaudages. Près de 40 millions d'euros auraient déjà été avancés à l'État avant le versement versement des premiers dons. Le projet annuel de performances pour 2020 n'indique pas la ligne de crédits sur laquelle cette somme a été prélevée ni les modalités de sa réaffectation vers d'autres projets. Je rappelle que 922 millions d'euros de promesses de dons ont été enregistrés, 67 millions d'euros ayant déjà été versés à l'État. L'établissement public administratif chargé de la restauration et de la conservation de la cathédrale vient, quant à lui, d'entrer en fonction. L'intégralité de son budget serait couverte par les dons. Or je vous rappelle, monsieur le ministre, que vous vous étiez engagé ici même au Sénat sur une participation de l'État. Vous aviez en effet indiqué que l'État devrait prendre sa part au financement de la restauration de Notre-Dame de Paris et qu'il y aurait, quoi qu'il en soit, des subventions budgétaires du ministère de la culture à l'établissement public. Quelques mois plus tard, il ne reste rien de cette volonté dans le présent projet de loi de finances. Une telle évolution rend indispensable la recherche de financements alternatifs, qu'il s'agisse du loto du patrimoine ou de dispositifs fiscaux spécifiques. La faiblesse des crédits budgétaires alloués à la restauration des centres-villes rend

Cette somme est à comparer aux 338 millions d'euros prévus dans le projet de loi de finances pour l'entretien et la restauration des monuments historiques. Nous appuyons les conclusions de conclusions de l'inspection générale des affaires culturelles et de l'inspection générale des finances qui vont dans ce sens. Nous invitons à proroger le mécanisme et à simplifier les conditions d'utilisation

Je suis par ailleurs inquiet du mauvais signal envoyé au travers de la réforme du mécénat d'entreprise, prévue dans le présent projet de loi de finances. Cette réforme a suscité une inquiétude légitime dans le milieu associatif, mais aussi au sein des organismes culturels, dont une partie de l'activité dépend du mécénat. Soyons clairs, le mécénat n'est pas une véritable niche fiscale. Le don vient parfois compléter, voire se substitue à l'action de l'État dans un contexte de réduction des marges de manoeuvre budgétaires de celui-ci. Le cas est particulièrement patent pour les opérateurs publics. L'État conditionne la reconduction ou une diminution minimale des subventions à des résultats sur divers critères d'ordre artistique, qualitatif, social ou sociétal, à propos de chantiers pour lesquels le soutien du mécénat est primordial. Les travaux d'ampleur menés pour le Grand Palais, la Cité du théâtre ou l'aménagement de l'Opéra Bastille s'appuient d'ailleurs sur le mécénat à la demande de l'État. Il existe donc une forme de schizophrénie de la part du Gouvernement dans le fait d'inciter les opérateurs publics à recourir au mécénat tout en limitant le plein et parfait développement de celui-ci. Le seuil de 2 millions d'euros au-delà duquel le taux de réduction passerait de 60 à 40 % peut paraître tout à la fois contournable et fragilisant. Dans tous les cas, le signal négatif envoyé par une telle réforme est bien tangible. Celle-ci laisse en effet entendre que toute opération dont le coût est supérieur à 2 millions d'euros est assimilable à une forme d'optimisation fiscale. Elle pourrait donc brider les intentions des mécènes, qui prendraient un risque en termes d'image. Nous savons que le Gouvernement a lancé une réflexion générale sur la philanthropie, qu'il a confiée à deux députées. Il aurait sans doute fallu attendre les conclusions de nos collègues sur les contreparties ou le régime juridique des fondations avant de procéder à

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « le patrimoine doit être une grande cause nationale » :ce n'est pas seulement le voeu de la commission de la culture, et du Sénat dans son ensemble ce sont les mots du Président de la République, Emmanuel Macron, lors du lancement du loto du patrimoine le 31 mai 2018. le niveau des crédits et développer de nouveaux instruments financiers en faveur du patrimoine monumental. Je pense en particulier au loto du patrimoine, qui en est maintenant à sa deuxième édition, et au fonds incitatif et partenarial pour la restauration des monuments historiques des petites communes à faibles ressources, qui permet d'impliquer progressivement les régions dans l'exercice des compétences en matière patrimoniale. Les ressources que procurent ces deux instruments restent, malgré tout, relativement modestes. Attention, dans ces conditions, à ne pas reprendre d'un côté ce qui est donné de l'autre ! Je ne vous le cache pas, monsieur le ministre, les signaux d'alarme ne manquent pas à cet égard, et j'en citerai deux. la réduction de 7 millions d'euros des crédits octroyés par l'État pour la restauration des monuments appartenant aux collectivités territoriales ou aux personnes privées, malgré leurs évidents besoins d'accompagnement.

La suppression de la réserve parlementaire en 2017 a déjà eu des effets dramatiques. Imaginez que cette réforme vienne purement et simplement casser la dynamique positive lancée par la mission Bern J'ajoute qu'elle est assez contradictoire avec l'obligation imposée aux opérateurs d'accroître leurs ressources propres et avec la décision de relever exceptionnellement le taux de défiscalisation pour financer la restauration de Notre-Dame Notre-Dame, justement ! Vous ne serez pas surpris, monsieur le ministre, que nous déplorions que l'État ne dépense pas un euro pour sa restauration, alors que nous avions clairement indiqué, au printemps dernier, lors du débat dans cet hémicycle, qu'il n'était pas acceptable que les coûts de fonctionnement de l'établissement public soient couverts par le produit des dons. Nous espérions au moins que l'élan de générosité aurait libéré des crédits en faveur des autres monuments, notamment de nos autres cathédrales. Très bien ! Nous constatons à regret que tel n'est pas le cas. Vous avez même envisagé d'annuler plus de 20 millions d'euros dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2019. C'est la preuve que des efforts doivent être poursuivis, afin d'améliorer la consommation des crédits : il est clair qu'elle ne trouve pas son origine dans un manque de besoins Néanmoins, compte tenu de la légère hausse enregistrée par ceux-ci, la commission de la culture a donné un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 175, « Patrimoines », et sera particulièrement attentive aux conséquences des évolutions envisagées sur la protection de notre patrimoine.

pour avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est difficile de porter un jugement tranché sur le budget pour 2020 pour deux des programmes de la mission « Culture » : les programmes 131 et 224. Dans les grandes masses, les crédits d'intervention destinés à la création sont préservés, comme les crédits dédiés à l'accès à la culture et à l'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministère de la culture. Mais c'est non sans sacrifices ! Crédits d'investissement, fonds de roulement des établissements, tout y passe ... au risque de voir bientôt disparaître toute marge de manoeuvre ! Je ne vous cache pas, monsieur le ministre, que cette stratégie nous inquiète, car elle nous paraît difficilement soutenable. C'est la deuxième année consécutive que vous la mettez en oeuvre et nous voyons mal comment vous parviendrez à la reconduire une troisième fois. Sans compter qu'elle renforce la crainte d'un désengagement progressif de l'État vers les collectivités territoriales ou les acteurs privés. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans quelques mois lors de l'examen du projet de loi « 3D », mais reconnaissez que les appels aux collectivités se multiplient pour qu'elles mettent en oeuvre et, surtout, financent les grandes priorités nationales : le pass culture, les Micro-folies et (EAC). C'est sans doute la seconde difficulté de ce budget : comment juger, à ce stade, de la pertinence de certains outils captant une part croissante des crédits, au détriment des politiques jugées plus structurelles ? Je pense, en particulier, au pass culture, qui pourrait être doté de 49 millions d'euros l'an prochain, alors que les crédits destinés à l'EAC, en tant que telle, sont en baisse et ne représentent même pas le double de ces crédits : 96 millions d'euros. Les premiers résultats de l'expérimentation, parus voilà deux semaines, sont mitigés et ne démontrent pas encore que le pass culture permettra de réduire les inégalités sociales et territoriales faisant obstacle à l'accès des jeunes à la culture, ou même de diversifier leurs pratiques

N'oublions pas non plus qu'à la base de toute politique culturelle il y a d'abord des artistes et des oeuvres. Attention donc à ne point assécher les crédits destinés à la création et à la structuration de ce secteur,

elle a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Culture

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà soixante ans était fondé le ministère de la culture. Créé pour et par André Malraux, son premier et seul ministre d'État, sa mission était, pour l'auteur de et de, « de rendre accessibles les oeuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des oeuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent L'année suivante, en 1960, était inaugurée la première maison de la culture à Béthune, puis celle du Havre, en 1961. À cette occasion, André Malraux rappelait que le IV plan en prévoyait la constitution d'une vingtaine dans les quatre ans. Il résumait ainsi son ambition Il s'agit de faire ce que la III République avait réalisé, dans sa volonté républicaine, pour l'enseignement ; il s'agit de faire en sorte que chaque enfant de France puisse avoir droit aux tableaux, au théâtre, au cinéma, etc., comme il a droit à l'alphabet Défendant son budget devant le Parlement en octobre 1966, il ajoutait : « Religion en moins, les maisons de la culture sont les modernes cathédrales : le lieu où les gens se rencontrent pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en eux. Sachez que chaque fois que nous en bâtissons une dans une ville moyenne, nous changeons quelque chose d'essentiel en France. » Soixante ans après, que reste-t-il de cette ambition ? Le pass culture ? Ce dispositif nous semble symptomatique de la perte de sens des politiques soutenues par le ministère de la culture. Les rares données disponibles pour l'expérimentation en cours laissent à penser que ce dispositif n'a pas favorisé la diversification des pratiques culturelles, mais, au contraire, qu'il a conforté les jeunes dans leurs choix actuels, échouant à intéresser à la culture les adolescents qui en sont les plus éloignés. Avec la rapporteure pour avis, Sylvie Robert, nous considérons qu'une politique publique dans le domaine de la culture doit nécessairement mettre à profit et contribuer à développer le réseau des structures culturelles et, plus particulièrement, celles qui sont aidées ou gérées par les collectivités locales. À l'opposé, le pass culture, promu par une société privée, risque de renforcer encore davantage l'emprise des plateformes qui captent déjà une grande partie de l'offre culturelle. Les capacités d'intervention de l'État s'en trouveront réduites. Enfin, nous regrettons vivement que la montée en puissance rapide et peu contrôlée du pass culture menace l'existence même de l'éducation artistique et culturelle. Il est encore temps de suspendre cette expérimentation pour délivrer aux jeunes un autre message : éteignez vos portables et, selon la formule d'André Malraux, allez à la rencontre des gens pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en vous Le choix politique de confier les missions de l'État à des entités constituées à l'extérieur du cadre de ses administrations a présidé, de la même façon, à l'organisation du chantier de sauvetage et de restauration de la cathédrale Notre-Dame En juillet dernier, des engagements avaient été pris dans cet hémicycle pour que l'État contribue à son financement. Las ! Nous apprenons aujourd'hui que l'établissement chargé de la conservation disposera d'un budget alimenté en totalité par les dons privés et que ses compétences exclusives en feront l'unique régisseur de toutes les interventions sur le monument. Comme je le craignais, ce chantier bénéficie ainsi d'une forme d'extraterritorialité, le constituant de fait en une petite principauté insulaire placée sous la seule autorité d'un coprince et aux frontières martialement défendues À la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, le ministère de la culture a heureusement décidé d'un plan de rénovation des systèmes de protection contre l'incendie dans les 89 édifices de culte dont il est propriétaire. plan sera mis en oeuvre par tous les acteurs du patrimoine- l'on regrette qu'une collaboration similaire n'ait pas été retenue à Paris. Il est doté d'un budget de 2 millions d'euros en 2020. Le rapporteur spécial vient de souligner, très justement, que cette mobilisation budgétaire a été réalisée aux dépens des crédits destinés aux opérations de restauration des monuments appartenant aux collectivités et aux propriétaires privés. Nous regrettons avec lui ce transfert, qui s'inscrit malheureusement dans un revirement majeur des choix politiques ministériels, dont témoignent aussi la faiblesse des moyens consacrés au patrimoine des centres anciens ou l'obsolescence programmée du dispositif fiscal dit Malraux. Dans ce domaine aussi, le succès relatif du loto du patrimoine ne pourra remédier au désengagement de l'État dans des politiques patrimoniales structurantes conduites avec les collectivités. De révision générale des politiques publiques en modernisation de l'action publique, les missions du ministère de la culture ont profondément évolué et votre proposition de budget pour l'année 2020, monsieur le ministre, Il devient urgent d'en tirer toutes les conséquences politiques et de procéder à un examen sincère de la place et du rôle du ministère de la culture, soixante ans après sa création. La parole

le ministère de la culture fêtait cette année son soixantième anniversaire. Depuis sa création sous l'égide d'André Malraux, le fil conducteur de son action n'a cessé d'être l'accessibilité de la culture pour tous.

rassemble les crédits destinés à financer les trois priorités de notre politique culturelle : le patrimoine ; la création ; la transmission des savoirs et la démocratisation de la culture. J'évoquerai en premier lieu le pass culture, qui bénéficiera de 10 millions d'euros supplémentaires pour financer son développement. L'initiative est heureuse eu égard à ses objectifs. Nous espérons qu'elle sera en mesure de s'adapter à l'ensemble des réalités territoriales. Les territoires bénéficieront de la création d'un réseau de 1 000 Micro-folies à l'horizon de 2022. Ces nouveaux musées numériques de proximité, qui ont vocation à s'implanter dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais également en milieu rural,

Ces nouveaux moyens permettront d'amplifier les aides accordées aux collectivités locales pour accompagner la création de nouvelles structures, diversifier leurs activités et étendre les horaires d'ouverture. Ce plan est également très apprécié dans les territoires. Le projet Démos sera doté de 2 millions d'euros et contribuera à diffuser la pratique musicale en zone rurale et au sein des quartiers prioritaires. La musique n'est pas l'apanage d'une élite issue des grandes villes. Le grand compositeur et violoniste George Enesco était fils d'agriculteur. Je pourrais citer le jeune Mourad, prodige des quartiers nord de Marseille, découvert alors qu'il jouait sur le piano du hall d'attente de l'hôpital de la Timone. Favoriser l'accès à la musique classique par la pratique instrumentale en orchestre est une belle initiative qui doit se développer. Enfin, nous saluons également la généralisation du dispositif d'éducation artistique et culturelle, doté l'an prochain d'un budget de 198 millions d'euros. L'année 2020 sera aussi marquée par de grands chantiers culturels : la rénovation du château de Villers-Cotterêts, symbole historique et futur berceau de la langue française, suit son cours dans les Hauts-de-France. La création d'une cité du théâtre représente un budget de 7 millions d'euros en 2020, sur un total de 86 millions d'euros d'investissement. Pour libérer les Ateliers Berthier, qui accueilleront cet espace, le Gouvernement prévoit la création d'une nouvelle salle modulable au sein de l'Opéra Bastille, dont le budget s'élève à 59 millions d'euros. Par ailleurs, le Centre national des arts plastiques se verra relocalisé sur le site de Pantin. Si les travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris seront entièrement financés par l'argent collecté lors de la campagne de souscription publique, le Gouvernement prévoit de consacrer 2 millions d'euros au plan d'action « sécurité cathédrales Le fonds incitatif et partenarial pour la restauration des monuments historiques des petites communes à faibles ressources bénéficiera de 10 millions d'euros l'année prochaine. En contrepartie, un effort particulier sera demandé au musée du Louvre, dont la dotation accusera une baisse de 15 %. L'autre versant, souvent négligé de nos politiques culturelles, et pourtant condition de leur existence, consiste au soutien à la création artistique, au sein du programme 131. Les crédits soutenant le fonctionnement des labels et des structures hors labels seront légèrement revalorisés et le spectacle vivant bénéficiera d'un effort particulier. Nous insistons sur la nécessité de sécuriser les parcours professionnels des artistes en développant les possibilités de résidence et en contrôlant davantage les rémunérations. Plus globalement, ces trois programmes s'inscrivent dans un double mouvement de déconcentration et de décentralisation des politiques culturelles. D'une part, l'administration centrale sera déchargée l'année prochaine de la gestion de 63 dispositifs au profit des DRAC. Pour accompagner ces transferts, nous saluons la création de 20 équivalents temps plein au sein de ces DRAC. D'autre part, l'année 2020 sera marquée par l'affirmation du rôle des collectivités locales dans le développement des projets culturels locaux, invitant l'État à repenser les termes du dialogue avec la mise en place du Conseil des territoires pour la culture. Nous saluons également la création prochaine d'un nouveau volet culturel au sein des futurs contrats de plan État-région. Nous sommes plus réservés sur l'article 50 du PLF prévoyant de diminuer le taux de réduction d'impôt en faveur du mécénat pour les plus grands donateurs. Nous soutenons fortement, en revanche, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en faveur du développement du mécénat de proximité, à savoir la relève de la franchise du plafond de 0,5 % du chiffre d'affaires instaurée par la loi de finances pour 2019, avec un nouveau plafond de 20 000 euros. Cette mesure devrait contribuer à favoriser l'engagement des PME et TPE dans le financement de projets

Tout d'abord, reposons ce postulat : une politique culturelle nationale ne saurait se faire au détriment des politiques locales et, inversement, les politiques locales ne sauraient exister sans une politique nationale portant une véritable vision. Même constat à propos de la politique patrimoniale. Tout patrimoine, classé, inscrit ou non, grand monument historique ou petit patrimoine vernaculaire, participe d'un ensemble cohérent, méritant une égale attention de l'État.

Quant aux Micro-folies, si là où elles sont installées les bénéfices sont visibles, leur modèle reste aussi fragile, car fonctionnement et médiation sont à la charge des collectivités. Pour une commune rurale, c'est extrêmement lourd

Le plan Conservatoires, bien qu'annoncé depuis deux ans, n'a toujours pas abouti. Quant aux crédits déconcentrés, leur déclinaison locale reste encore l'objet de fortes disparités. Nous attendons les propositions du ministère pour une répartition plus juste et adaptée aux besoins sur le territoire national. Sans critères véritablement formalisés et sans orientations claires, les collectivités locales, pour le moment, ne voient pas venir cette liberté tant attendue. Les DRAC ont peu de souplesse. Une fois les obligations budgétaires assumées, difficile de trouver des reliquats de crédits en soutien aux initiatives locales, certes atypiques

Ces actions reposent beaucoup sur la bonne volonté de l'établissement scolaire et des collectivités, qui en sont les grands financeurs. Monsieur le ministre, nous attendons vraiment le contenu du travail interministériel entre l'éducation nationale et la culture. Cet Objectif 100 % éducation artistique et

Pour le budget du patrimoine, nous pouvons faire le même constat, celui d'un délicat équilibre entre le national et le local. Le budget pour 2020 est en légère hausse, c'est une très bonne nouvelle. Mais, dans sa déclinaison territoriale, cette augmentation est inégalement répartie. Vous le savez, une forte injustice est ressentie entre les grands travaux parisiens et la province. Si l'effort réel consenti en direction du patrimoine monumental est présenté comme le fruit d'économies sur le musée du Louvre, il y a aussi, en réalité, des redéploiements de crédits. En particulier, une diminution de l'ordre de 5 % des subventions d'investissement accordées aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés en vue de la restauration de monuments historiques. Ces derniers disposent pourtant du plus grand nombre de monuments en péril. La question de la conservation de ceux-ci est de nouveau posée. Nous soutiendrons donc l'amendement de la commission des finances sur le sujet. Le patrimoine vernaculaire, certes moins spectaculaire, se voit attribuer une mince partie du budget. Répétons qu'il fait l'âme des territoires et que les Français y sont attachés, comme l'a montré la mission Bern. Le patrimoine est un tout. Monument historique ou petit patrimoine, inscrit, classé ou non, l'État doit y veiller et avoir le souci de considérer chaque entité. À ce titre, la non-compensation des taxes du loto du patrimoine est à mettre au compte des mauvais signaux. La réforme, à l'article 50 du PLF, de l'avantage fiscal au bénéfice du grand mécénat fragilise cette ressource essentielle aux territoires. Ajoutons cette autre menace fiscale portant sur le dispositif Malraux. Ces messages sont déstabilisants. L'écosystème du patrimoine est délicat, avec une répartition, toujours sur une logique de crête, des financements entre le privé et le public. Il est fragilisé actuellement avec ces contradictions permanentes.

Enfin, hors la question des moyens, celles des besoins organisationnels, techniques et en termes d'expertise se posent. C'est pourquoi les DRAC doivent rester disponibles, auprès des territoires, pour le patrimoine. Reposons la question de la compétence de l'État en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle fait cruellement défaut Monsieur le ministre, je terminerai en insistant sur le rôle majeur joué pas les collectivités territoriales, qui, en France, restent les premiers financeurs de la culture et, pour une grande partie, du patrimoine. La perte de plus en plus grande de l'autonomie financière des collectivités a une forte Les acteurs du secteur sont inquiets, car, au fil des années, les budgets tendent vers d'impossibles équations et les dépenses culturelles et patrimoniales se réduisent déjà dans certaines collectivités. Patrimoine ou culture, on le voit bien, la France a besoin d'une politique territoriale et d'une politique nationale qui s'unissent et se complètent. Décentraliser et déconcentrer plus, cela signifie, aussi, assurer la cohérence nationale. L'État doit éviter les actions trop visibles ou communicantes et se consacrer surtout au travail laborieux et minutieux sur le terrain, aux côtés des collectivités, pour décliner avec justesse et justice l'accès à la culture, consacrant les droits culturels, d'une part, et la valorisation du patrimoine, de l'autre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits dédiés à la culture dans le PLF pour 2020 doivent contribuer à faire vivre une politique culturelle ambitieuse pour notre pays, mais ils restent sous le seuil symbolique de 1 % du budget global.

De plus, certaines actions s'appuient davantage sur les financements décentralisés des collectivités territoriales. Je note un autre point frappant : des lignes budgétaires n'ont pas été totalement consommées en 2019. C'est le cas pour l'expérimentation du pass culture, j'y reviendrai. En bref, le budget de la culture est cette année encore contrasté. Si une baisse de 3,36 % des autorisations d'engagement de la mission est prévue, les crédits de paiement connaissent une légère hausse de 2,93 à 2,95 milliards d'euros. Ces chiffres traduisent une relative stabilité, qui cache des situations contrastées. Les principaux axes de ce budget sont le soutien à l'emploi culturel, le développement de l'expérimentation du pass culture et la poursuite de grands travaux- Versailles, le Grand Palais, ou encore Villers-Cotterêts -, dotés de 30 millions d'euros, issus du programme d'investissements d'avenir et des crédits destinés aux monuments historiques, pour les grands projets. Les faibles moyens alloués à la restauration des centres-villes dans le cadre du plan Action coeur de ville, soit seulement 8,9 millions d'euros pour 880 sites patrimoniaux remarquables répertoriés, traduisent un manque d'ambition, unanimement regretté au sein du groupe RDSE, beaucoup restant une fois de plus à la charge des communes. En outre, à la suite du dramatique incendie de Notre-Dame de Paris, de savants jeux d'écriture font passer des crédits prévus pour les subventions destinées aux collectivités territoriales vers le financement de la sécurisation des cathédrales, pour un montant de affectant injustement les collectivités. En 2019, je faisais déjà part de mon scepticisme face au loto du patrimoine. Pour cette deuxième édition, étant donné son succès auprès de la population, cette opération devrait rapporter des gains prévisionnels estimés à 25 millions d'euros au moins.

Ce type d'initiative laisse croire que l'on peut se satisfaire d'opérations ponctuelles pour mener des actions d'entretien du patrimoine, qui fait la richesse de notre pays. La multiplication d'opérations de cette nature ne peut se substituer à l'action publique sans avoir de conséquences à long terme. Pour atteindre le but visé, il aurait été plus efficace d'encourager nos concitoyens à effectuer des dons directement auprès des associations de gestion du patrimoine. Cette question reste entière, et je garde un avis personnel J'en viens au programme 224, « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », dédié notamment aux politiques transversales d'éducation artistique et culturelle, dont les crédits de paiement progressent, à périmètre constant, s'établissant à 1,17 milliard d'euros en 2020. englobe le déploiement, à l'horizon 2022, d'un millier de Micro-folies, mini-musées numériques de proximité, pour 3 millions d'euros. Ces structures sont censées faciliter l'accès de tous aux grandes oeuvres de notre patrimoine. Toutefois, leurs coûts de fonctionnement et de maintenance seront, encore, à la charge des collectivités locales. L'effort consacré à l'expérimentation du pass culture, en hausse de 35 %, atteignant 39 millions d'euros, semble se faire au détriment des crédits pour l'éducation artistique et culturelle qui, hors pass culture, sont en baisse, comme l'a relevé la rapporteure pour avis. À plein régime, ce dispositif mobilisera 400 millions d'euros ; c'est autant d'argent public qui doit être utilisé à bon escient, et pas seulement dans l'intérêt économique des prestataires culturels. Permettra-t-il d'atteindre l'objectif affiché de pérenniser à long terme l'appétence culturelle de nos jeunes et leur accès à la culture ? Nous aimerions disposer d'un bilan scientifique plus précis de l'incidence réelle de cet effort financier sur la réduction des barrières sociales et territoriales d'accès à la culture. Présidente du groupe d'études Arts de la scène, arts de la rue et festivals en région, j'évoquerai encore deux points. Tout d'abord, les problèmes de sécurisation des festivals n'ont pas disparu, au contraire, et les coûts ont augmenté depuis la publication de la circulaire Collomb. Cette question nécessitera sans aucun doute une évaluation dans le cadre du nouveau fonds d'intervention pour la sécurité des manifestations culturelles et la sécurité des sites de presse, créé par le décret du 18 mars 2019. des précisions sur la consommation des crédits de ce fonds depuis sa mise en place seraient effectivement bienvenues, pour procéder à un état des lieux budgétaire. En outre, je rappelle mon attachement à la pérennisation des crédits d'impôt dans le secteur culturel, car ils sont bénéfiques à la diversité et à la création d'emplois.

plus amples précisions de votre part, monsieur le ministre, le groupe RDSE votera les crédits de la mission « Culture ». La parole

En conséquence, nombre des moyens nouveaux n'opèrent qu'un retour en arrière et compensent simplement les baisses de ressources des années passées. L'ensemble reste cependant satisfaisant dans le contexte actuel de maîtrise des dépenses publiques, comme l'ont souligné les rapporteurs. Je ne détaillerai pas l'ensemble des crédits, mais je souhaite évoquer plusieurs sujets d'inquiétude. Je commencerai par le patrimoine. Le terrible incendie de Notre-Dame de Paris a mis en lumière le manque de moyens alloués à la préservation des monuments historiques, notamment de nos édifices religieux.

Ainsi, 23 % des immeubles protégés au titre des monuments historiques sont en mauvais état, et près de 5 % en situation de péril. Les annonces traduisent donc plus un affichage politique qu'un réel investissement. Je veux également souligner le paradoxe que connaît cette année le mécénat. Au fil du temps, le mécénat est devenu le mode de financement naturel des institutions culturelles et de la rénovation de nos monuments historiques. En 2020, l'État compte plus que jamais sur lui, qu'il s'agisse de la rénovation de Notre-Dame de Paris, mais aussi d'autres grands chantiers, tels que tels que celui du château de Villers-Cotterêts, où un apport de 25 millions d'euros est attendu, soit près d'un quart du budget total du projet. L'État encourage d'ailleurs ses grands opérateurs à attirer des mécènes, ce qu'ils font avec succès. par l'article 50 du PLF que nous examinerons prochainement, le Gouvernement souhaite durcir la fiscalité du mécénat, en diminuant de 60 % à 40 % la réduction d'impôt pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros. Aucune étude d'impact n'a été réalisée en amont. De plus, cette réforme intervient alors que le Premier ministre a confié à deux députées une mission visant au développement de la philanthropie française. Comment expliquer alors que le Gouvernement, au nom de la rigueur fiscale, prenne le risque de porter préjudice au mécénat ? Mon groupe soutiendra bien évidemment les initiatives revenant sur cette disposition. Je souhaite dire également quelques mots sur l'objectif fixé par le Gouvernement d'un égal accès de 100 % des jeunes aux arts et à la culture. L'émiettement des crédits consacrés à l'éducation artistique et culturelle reflète les contours flous de ce projet. Les financements se concentrent surtout sur la mesure phare du pass culture, promesse de campagne, certes séduisante, du Président de la République. Cette enveloppe de 500 euros destinée aux jeunes de 18 ans, mise en place pour le moment dans 14 départements, vise à terme tous les jeunes résidant en France. Le PLF anticipe une montée en charge de ce dispositif,

Le pass culture ne saurait être le seul vecteur utilisé pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales, et son développement ne doit pas s'opérer au détriment des actions traditionnelles. Je crains surtout que ce projet ne soit peu réaliste. La première expérience en la matière a en effet été un échec. Le italien a donné lieu à des trafics en tout genre : reventes de livres, émissions de fausses factures, achats de produits américains ou sud-coréens, etc. Le dispositif mis en place pourra-t-il éviter ces mêmes dérives ? L'autre écueil serait que le pass culture manque son public. Le n'a profité qu'à la moitié des jeunes, précisément ceux qui avaient déjà accès à la culture. C'est dommage Les premières données de l'évaluation conduite sur le pass culture sont peu encourageantes, avec un taux d'activation de seulement 52 %, et un taux d'utilisation parmi les jeunes ayant créé un compte de 68 %. %. C'est surtout le profil exact des bénéficiaires qu'il faudrait connaître, avant d'envisager une généralisation du dispositif à toute la France. Par ailleurs, il me semble que cet effort important de l'État serait plus utile s'il intervenait plus en dans la construction du jeune. Attendre l'âge de 18 ans est en effet bien tard pour sensibiliser un enfant à la culture. Je pense que cette ouverture pourrait et devrait d'abord se faire avec les instituteurs et les professeurs, au sein de l'école de la République, qui a pour mission l'éveil intellectuel de tous les élèves, sur l'ensemble du territoire. Nous serions ainsi certains de toucher tous les publics.

de la première maison de la culture inaugurée en 1961 par André Malraux dans la belle ville du Havre à aujourd'hui, quel chemin parcouru ! Sans nul doute, le ministère de la culture peut être un motif de fierté. Cependant, sa tâche est encore immense. Les défis que représentent l'accès à la culture pour toutes et tous, l'accès aux oeuvres et aux artistes, mais aussi l'accès à la pratique et les conditions de son exercice, les droits d'auteur, le statut des intermittents du spectacle, le patrimoine et les archives constituent les fondements de l'action du ministère. Par son expertise, son expérience et la grande qualité de ses agents, celui-ci a un rôle prépondérant à jouer dans le rayonnement culturel de la France et de ses territoires. il existe un paradoxe surprenant : la culture, produit d'une histoire mouvementée, fondée sur les expériences douloureuses de l'esclavage et de la colonisation, est foisonnante et plurielle, mais nous constatons dans le même temps les manques d'une politique culturelle qui, trop longtemps, a traité les outre-mer en parents pauvres. Comme le montrait en 2018 le rapport sur les zones blanches de la culture, il reste beaucoup à accomplir pour réduire les inégalités patentes qui demeurent entre les différents territoires de l'Hexagone, et entre l'Hexagone et les outre-mer. et les outre-mer. Trente-sept ans après le premier mouvement de décentralisation culturelle des lois Auroux, les chiffres révèlent un sous-équipement flagrant. Pour les 2,7 millions d'Ultramarins répartis dans une dizaine de territoires, au total seulement deux conservatoires et deux scènes nationales, aucune salle de plus de 3 000 places, aucun musée d'art contemporain et un seul fonds régional d'art contemporain (FRAC) situé sur l'île de la Réunion. Il faut le dire, longtemps le pouvoir jacobin a nié nos spécificités culturelles, craignant de nourrir des velléités indépendantistes.

Toutes ces missions appellent à renforcer les services déconcentrés de l'État, à associer les collectivités territoriales, à conforter les associations et à s'appuyer avec cohérence sur les groupes privés. Il faut les renforcer à travers une politique ambitieuse et ouverte à la création, une politique de soutien à toutes les actrices et à tous les acteurs de la culture. Comme ces deux dernières années, les crédits de la mission « Culture » sont maintenus en 2020, avec une hausse de 1 % par rapport à la loi de finances pour 2019. Le budget qui nous est présenté se veut d'abord au service de l'émancipation citoyenne. Pour cela, vous engagez,

présenterons dans quelques jours le fruit de notre travail sur les nouveaux territoires de la culture. Nous défendrons notamment l'urgence de combattre les inégalités territoriales- elle l'a signalé il y a quelques instants -, que j'ai décrites précédemment, au profit d'un nouveau modèle de démocratisation culturelle fondé sur la notion de droits culturels. L'émancipation citoyenne passe également par le pass culture. Pour observer l'expérimentation à l'oeuvre sur mon territoire et participer à son suivi au sein du groupe de travail présidé par Jean-Raymond Hugonet, je peux témoigner de l'investissement des services déconcentrés de l'État et des effets déjà bénéfiques de ce dispositif. En 2019, une nouvelle étape a été franchie avec la poursuite de l'expérimentation et le lancement de la société du pass culture. L'an prochain, 10 millions d'euros supplémentaires, soit un total de près de 40 millions d'euros, nous permettront d'accroître le nombre de jeunes éligibles et d'ouvrir l'expérimentation à de nouveaux territoires. Cela étant, les résultats de la première expérimentation montrent que 52 % des jeunes auraient activé leur compte. Peut-être pourrez-vous nous dire, monsieur le ministre, les moyens que votre ministère entend mettre en oeuvre pour que les jeunes aient une meilleure connaissance du dispositif lors des expérimentations à venir. Les crédits alloués au programme « Création » sont, eux aussi, en augmentation. Le spectacle vivant se trouve ainsi renforcé à travers, entre autres, les grands opérateurs, importants vecteurs culturels irriguant le territoire ils sont des acteurs essentiels qui participent à la transmission des savoirs au plus grand nombre. Je salue l'initiative des Micro-folies, opportunités formidables de diffusion de la culture. outre-mer, ce dispositif a été lancé avec succès, le 16 novembre dernier, en Guadeloupe, avec l'inauguration des deux premières Micro-folies, dont une itinérante sur l'ensemble du territoire. Enfin, les crédits du programme 175, « Patrimoines », de la mission « Culture » progressent de 6,8 %. Les 970 millions d'euros du programme sont, pour une large part, dévolus à l'entretien et à la restauration des monuments historiques et du patrimoine monumental, avec quelques chantiers particulièrement importants, comme le Grand Palais à Paris ou le château de Villers-Cotterêts. Ce château, méconnu de la plupart des Français, fait partie des hauts lieux de l'histoire de France. Il accueillera un projet francophone unique au monde, la cité internationale de la langue française, auquel nous adhérons tous- je suppose -sur ces travées. l'année 2019 a été marquée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le fonds dédié à la mise en oeuvre du plan de sécurisation des cathédrales, doté de 2 millions d'euros, doit financer des audits qui nous permettront de nous assurer qu'une telle catastrophe ne frappe jamais l'une des 87 cathédrales classées appartenant à l'État. Si ces chantiers sont évidemment indispensables, nous sommes heureux de constater que le budget alloué aux patrimoines de moindre ampleur est lui aussi en augmentation. Il est nécessaire d'envoyer, à l'adresse des collectivités, un signal pour montrer que l'État réinvestit dans ce patrimoine, qui est tout aussi important. Nous savons toutefois que les chantiers, en ce domaine, sont multiples et pratiquement inépuisables ; c'est pourquoi l'effort devra être prolongé. le budget de la présente mission progresse ; il va dans le sens d'une meilleure prise en compte de tous les territoires et privilégie les structures souples, qui s'adressent en priorité aux plus jeunes de nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, mon groupe votera les crédits de la mission « Culture

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous célébrons les soixante ans du ministère de la culture, il paraît opportun de rappeler l'ampleur de la mission assignée par son décret fondateur : « rendre accessibles premier objectif de rendre accessibles les oeuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser oeuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent ». Le présent budget est-il à la hauteur de ces enjeux primordiaux ? Vous vous félicitez, monsieur le ministre, de nous présenter un budget ambitieux, en hausse de 73 millions d'euros,

Au sein du programme « Création » a été créée l'action n° 06, Soutien à l'emploi et structurations des professions, par transfert de l'action n° 08 Dotée de 38 millions d'euros, elle bénéficiera notamment au Fonpeps. Celui-ci a fait l'objet d'une refonte, mise en oeuvre le 1 octobre dernier : une aide unique à l'embauche en CDI en CDD se substitue aux quatre premières mesures du fonds initial. Nous souhaitons que cette restructuration permette une plus grande lisibilité et une meilleure efficacité du dispositif. En outre, nous saluons le maintien de la compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), qui avait entraîné une baisse du pouvoir d'achat des artistes-auteurs. Nous resterons vigilants sur la mise en oeuvre de la vaste réforme du statut social des professionnels du secteur. Au sein du programme 224, l'action n° 01, Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle, connaît cette année encore une baisse de 5 millions d'euros ; l'érosion des crédits de cette action se poursuit. Sans artiste, monsieur le ministre, pas de culture ! Un effort budgétaire plus important doit être consenti, afin de préserver la qualité des formations et de favoriser l'accompagnement des artistes vers la vie active : seuls 10 % des élèves diplômés parviennent à vivre exclusivement de leur pratique artistique ! De même, la révision du statut des professeurs des écoles d'art territoriales ne peut plus attendre. L'action n° 02, qui finance le soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle, est en légère hausse ; elle est consacrée en réalité au pass culture, dont l'enveloppe est portée à 39 millions d'euros. L'expérimentation se poursuit, notamment dans ma région, où 18 000 jeunes sont inscrits. Une mission d'évaluation est en cours et nous

monsieur le ministre, les jeunes utilisateurs ont souligné des dysfonctionnements de l'application et l'insuffisance des offres locales, notamment dans les secteurs ruraux, dans lesquels la mobilité est une question cruciale. Les professionnels s'inquiètent du manque de visibilité pour les petites structures. Nous demeurons vigilants à l'égard des déterminismes sociaux, géographiques et culturels, qui pourraient faire passer ce dispositif à côté de son objectif initial. La mise en oeuvre d'une véritable médiation paraît plus que nécessaire. Quant au mécénat, il a été évoqué à plusieurs reprises. Je n'y reviens pas. Pour conclure, nous regrettons le peu de références aux droits culturels, introduits dans la loi droits culturels doivent pourtant constituer le fil directeur de l'ensemble des acteurs concourant aux politiques culturelles. également à dégager une cohérence d'ensemble aux politiques publiques soutenues par votre ministère. Ce dernier apparaît aujourd'hui comme affaibli, peinant à engager et piloter une politique culturelle structurée et structurante. Affaibli, le ministère l'est d'abord par les coupes budgétaires imposées par Bercy ; il l'est aussi par la place toujours plus prépondérante prépondérante du secteur privé, qui entraîne la culture dans une logique marchande et financière en vertu de son propre désengagement. Si la culture est bien une compétence partagée, si nous ne pouvons que saluer l'effort annoncé en faveur d'une plus large déconcentration, ainsi que le travail conjoint avec les collectivités, cet aspect ne doit pas constituer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le patrimoine est le bien commun de tous les Français. Il est notre mémoire collective, notre trésor national. Son entretien, sa sauvegarde, sa mise en valeur sont une nécessité, un enjeu culturel éminent auquel il ne faut déroger en aucune façon, qu'il s'agisse du majestueux château de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, ou ou de la petite église romane de Châteauneuf-de-Bordette, dans les Baronnies provençales. Si cette année les crédits du programme 175 affichent une légère hausse en crédits de paiement- nous nous en réjouissons -, soulignons cependant que ce programme est « gonflé » de 63 millions d'euros supplémentaires provenant du programme 224. Hors transfert, le programme est en réalité en baisse de 1 % en crédits de paiement hors inflation. Ce budget, comme le soulignent les associations de protection du patrimoine, manque d'un certain élan, pourtant nécessaire pour concrétiser l'ambition que nous avons pour pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine dans tous les territoires. Le budget alloué à l'entretien et à la restauration des monuments historiques s'élève à 338 millions d'euros en crédits de paiement. Si les crédits destinés aux monuments historiques, hors grands projets, sont en légère hausse, atteignant 300 millions d'euros,

d'euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement est nécessaire pour permettre la restauration et l'entretien des monuments historiques. Le compte n'y est pas ! Le compte n'y est pas non plus pour les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), qui n'ont pas toujours les moyens d'aider les propriétaires à entretenir leur patrimoine. Beaucoup de collectivités et de propriétaires privés ont ont pourtant cruellement besoin d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO). Nous pensons d'ailleurs qu'un meilleur fonctionnement de l'AMO- la situation est très inégale selon les régions -permettrait sans doute d'améliorer la consommation des crédits chaque année. Il convient aussi, de la part du Gouvernement, de maintenir une certaine cohérence : on ne peut pas d'un côté afficher la protection du patrimoine comme un enjeu politique majeur en matière de culture, et d'un autre remettre en cause 25 millions d'euros de crédits en sa faveur dans le cadre du PLFR de 2019. Le Sénat- c'est tout à son honneur -a fort heureusement rétabli ces crédits. Concernant le loto du patrimoine, en adoptant, contre l'avis du Gouvernement, l'exonération des contributions à l'État, comme l'année dernière, le Sénat a une nouvelle fois été le gardien de la protection du patrimoine. Notre position est constante : l'État n'a pas à récupérer de nouvelles recettes sur ce loto. La totalité de l'enveloppe doit revenir au patrimoine, et non à Bercy. à Bercy. Par ailleurs, cette opération devrait être pérennisée, au-delà de 2020, même si, rappelons-le, ce type d'action doit avoir pour vocation de compléter et non de remplacer les subventions publiques. Il en va de même pour le mécénat. Le durcissement de la fiscalité que vous envisagez, aura évidemment des répercussions sur le financement du patrimoine ; il risque de casser une dynamique positive en sa faveur. Mon groupe a déposé un amendement, afin que le dispositif incitatif fiscal dont bénéficie grandement notre patrimoine ne soit pas modifié. J'espère que le Sénat aura la sagesse de l'adopter. Je ne peux parler de patrimoine sans évoquer le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Aucune ligne budgétaire n'est prévue. Le Gouvernement compte donc bien faire financer l'intégralité du chantier, y compris les coûts de fonctionnement de l'établissement public, par les donateurs privés, ce qui est pour le moins contradictoire avec vos propositions de réforme du mécénat, vous en conviendrez ! Voilà qui laisse un goût amer, face au désengagement de l'État vis-à-vis d'un chantier patrimonial emblématique.

Enfin, je dirai quelques mots du petit patrimoine rural, lequel est vital pour le rayonnement et le dynamisme de nos territoires. Je me réjouis de l'augmentation de 5 millions d'euros du fonds incitatif et partenarial

Depuis Malraux, l'ambition est la même : mettre la culture au centre de notre pacte social, en faire l'un des instruments privilégiés de la cohésion nationale, partout sur le territoire.

effort, qui nous impose des résultats. Or, pour obtenir des résultats, il faut établir des priorités. Le budget que je vous présente en dénombre quatre. Il est au service de l'émancipation de tous, au service de la cohésion et de l'attractivité des territoires, au service des artistes et des créateurs et, bien entendu, au service de notre souveraineté culturelle. La première priorité- l'émancipation des citoyennes et des citoyens -passe par la généralisation de l'éducation artistique et culturelle. La culture, c'est nous retrouver autour de ce que nous trouvons beau. C'est partager ce qui nous plaît, au sens le plus noble du terme. Mais encore faut-il pouvoir aller au-delà de ce que nous connaissons ; découvrir

la rencontre avec les oeuvres, comme la pratique d'une activité artistique, ne s'arrête pas à 18 ans. Elle s'étend tout au long de la vie. Chacun y a droit, quels que soient sa situation, son âge ou- j'y insiste -son lieu de vie.

Cette émancipation pour et par la culture, nous l'encourageons aussi par le pass culture, que nous concevons, pour les jeunes, comme un instrument de liberté

À l'origine, le pass culture est une belle idée : 500 euros à 18 ans pour accéder à des offres culturelles. Cette belle idée, nous sommes en train d'en faire une réalité. Nous mettons au point une application géolocalisée qui permet à chaque jeune d'accéder à l'offre culturelle située à proximité du lieu où il vit ou, tout simplement, du lieu où il est. En juin dernier, nous avons lancé une seconde vague d'expérimentation auprès de 150 000 jeunes. L'an prochain, 39 millions d'euros seront dédiés au pass culture, auxquels s'ajouteront 10 millions d'euros de reports de 2019 vers 2020, afin d'augmenter le nombre de jeunes éligibles- ils sont déjà plus de 35 000 -, d'ouvrir l'expérimentation à de nouveaux territoires et d'enrichir encore l'offre proposée.

Je sais que le groupe de travail présidé par Jean-Raymond Hugonet suit l'évolution de cette politique de très près. De plus, nous mesurons constamment la mobilisation des jeunes et des acteurs culturels. Cette mobilisation est capitale : c'est grâce à elle que le pass culture deviendra un outil de valorisation de l'offre culturelle dans nos territoires. La deuxième priorité de ce budget, c'est justement de renforcer la cohésion et l'attractivité de nos territoires. Nous les renforcerons d'abord par les services publics culturels de proximité. D'une certaine manière, il faut les conforter et les réinventer, en les adaptant aux nouvelles attentes de nos concitoyens dans un environnement marqué par l'irruption du numérique.

à l'action des collectivités locales, des acteurs culturels, des associations et, bien sûr, des artistes. Nos modes d'action doivent changer. Notre état d'esprit doit évoluer. En particulier, il faut déconcentrer les dispositifs de soutien déployés Une soixantaine d'entre eux seront concernés en 2020, dont la labellisation des centres culturels de rencontre et l'octroi des aides aux compagnies et aux festivals.

occasion pour saluer votre décision de maintenir la totalité des crédits de 2019 en faveur des patrimoines, au titre du projet de loi de finances rectificative. En 2020, près de 1 milliard d'euros seront consacrés aux politiques en faveur des patrimoines. J'ai le plaisir de vous confirmer que les moyens dédiés à l'entretien et à la restauration de nos monuments historiques augmenteront de 7 millions d'euros, pour atteindre 338 millions d'euros en crédits de paiement. Nous soutiendrons les investissements du Centre des monuments nationaux (CMN), qui, vous le savez, est un puissant outil d'égalité entre les territoires. Nous poursuivrons la montée en puissance du fonds incitatif et partenarial (FIP) en faveur des communes à faibles ressources. Par ailleurs- je le confirme -, nous financerons un plan de sécurité incendie pour les cathédrales classées appartenant à l'État.

dont Jean-Pierre Leleux a été le rapporteur, va elle aussi dans ce sens. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement l'a soutenue, en se prononçant pour le rehaussement du seuil des communes concernées par le label de la Fondation du patrimoine de 2 000 à 20 000 habitants. troisième priorité de ce budget est de placer les artistes et les créateurs au coeur de nos politiques culturelles. Je veux que les intéressés soient mieux accompagnés tout au long de leur parcours. Les dispositifs du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) ont été simplifiés et rendus plus incitatifs. En outre, les moyens Le dispositif de compensation de la hausse de la CSG pour les artistes-auteurs sera pérennisé. La politique de résidences sera réorientée et amplifiée. Accompagner les créateurs tout au long de leur parcours implique également de lutter contre leur précarité. S'engager dans l'art, dans la création, c'est effectivement prendre un risque : mais, cette prise de risque, nous en avons besoin,

Accompagner les créateurs suppose également de mettre à leur disposition des équipements adaptés. Nous poursuivrons le projet de Cité du théâtre. Nous mènerons à bien le projet de relogement, à Pantin, des réserves du Centre national des arts plastiques (CNAP) et du Mobilier national. Enfin, accompagner les artistes, c'est participer à la structuration des secteurs dans lesquels ils exercent. Là est tout l'enjeu de la création du Centre national de la musique. Cette maison commune de la musique verra le jour La quatrième et dernière priorité de ce budget est de réaffirmer notre souveraineté culturelle. C'est tout l'enjeu du projet de loi sur l'audiovisuel que j'ai présenté ce matin même en conseil des ministres

elle est notre héritage commun. Agissons, avec ambition, au service de tous les Français. Ce budget pour 2020- je veux le croire -nous permettra de favoriser leur émancipation, de soutenir la culture dans nos territoires, d'accompagner nos artistes et nos créateurs et, enfin, de réaffirmer notre souveraineté culturelle !

Monsieur le ministre,

du 18 mars. Ce fonds, comme vous le savez, succède au fonds d'urgence pour le spectacle vivant, qui a pris fin en décembre 2018. Les montants affectés au fonds d'urgence puis au fonds pérennisé ont connu une chute brutale, passant en 2019 à 2 millions d'euros. Cette somme, dont une partie est censée être utilisée pour la sécurité de certains acteurs de la presse, ne suffit pas. pas. L'année dernière, déjà, le Syndicat national du théâtre privé estimait les besoins à 1 million d'euros par an pour le théâtre et à 1,7 million d'euros pour le cabaret. Il faut ajouter à cela les besoins de tous les autres acteurs du spectacle vivant. La mission flash de l'Assemblée nationale sur les nouvelles charges en matière de sécurité pour les salles de spectacles et les festivals du 20 février dernier confirme d'ailleurs cette insuffisance des crédits. Nous vous proposons donc, par cet amendement, de rehausser le montant du Fonds d'intervention au son niveau du fonds

combien l'objet de cet amendement est important et alerter le ministre sur la sécurité et la sûreté des salles et des festivals. Tout s'est bien passé cette année, mais l'on sait que la circulaire Collomb

cet amendement tend à permettre la mise en place de moyens pour accompagner les cirques familiaux dans leur besoin de soutien et de développement. Quel

création. Des pôles nationaux du cirque sont chargés d'accompagner le secteur en termes de diffusion, de production et d'action culturelle. J'étais encore, il y a quelques mois, au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, qui assure la formation et l'insertion dans l'emploi des professionnels des arts du cirque. Mon ministère mène donc une politique ambitieuse d'accompagnement du cirque dans sa diversité. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur Leconte,

2020 ressemble, hélas !, à 2019. Nous restons dans la même logique d'application du programme d'économies imposé aux entreprises du secteur public de l'audiovisuel. Pourtant, rien ne justifie que les opérateurs de l'audiovisuel extérieur soient taxés parce que les autres le sont. Ce serait en effet nier leurs spécificités et leur importance, dont on se gratifie plus facilement dans les discours que dans les actes. Chacun s'alarme du regain des luttes d'influence sur les ondes et dans l'espace numérique ; chacun déplore la multiplication des actions de désinformation et de déstabilisation chacun s'émeut du développement des médias extérieurs par les États puissances, des restrictions portées à la liberté d'information et du maintien de la propagande des groupes terroristes sur internet et sur les réseaux sociaux chacun reconnaît qu'il est essentiel et de bon sens que la France puisse être présente et ne laisse pas à la merci de la propagande de nos adversaires des populations pour lesquelles elle engage, parfois, la vie de ses soldats- nous ne le savons que trop cruellement ! Chacun s'agite, Chacun s'agite, mais personne n'agit ! De cela découle notre agacement, voire notre vraie colère. Où est donc la cohérence entre les belles paroles au sommet de l'État, dans lesquelles nous nous reconnaissons, et les moyens comptés de nos opérateurs ?

stagne à 76,2 millions d'euros, alors que le plan stratégique appelait des financements plus importants. Ses objectifs de transformation numérique et de déploiement en Afrique auront été anticipés, mais ne pourront être entièrement Sa distribution sera réduite de 370 à 364 millions de foyers, avec l'abandon de la diffusion en Grande-Bretagne et en Irlande. En 2020, elle abandonnera le Brésil et l'Europe continentale, soit 32 millions de foyers en moins, ce qui aura une incidence sur son audience et sur ses ressources propres. Elle aura beaucoup de difficultés à financer la plateforme numérique de fictions francophones, initiée par le Canada, qui met au pot 9,5 millions d'euros, et à renouveler son outil de production et de diffusion. 12 millions d'euros sur quatre ans sont nécessaires. Il faudra encore restreindre la distribution et couper dans les programmes. La France est le seul pays à avoir réduit sa contribution depuis la création de TV5 Monde et ne respecte plus ses engagements. Cela ne la place pas dans une bonne situation au moment où un nouveau plan stratégique est en préparation. Les perspectives de France Médias Monde ne sont pas meilleures, hélas ! Ses crédits baissent de 1 million d'euros, alors qu'elle continue d'afficher de bons résultats d'audience en linéaire comme en numérique. Elle réalise les objectifs de son contrat : enrichissement des grilles de programme, ouverture d'un service en espagnol, adaptation aux évolutions des modes de diffusion ; elle produit, depuis cette année, un très important programme diffusé mandingue, indispensable dans une zone où nos armées sont engagées. Pour financer les impasses budgétaires, après avoir raclé les fonds de tiroir, elle est toutefois contrainte d'allonger la programmation à l'antenne des grilles d'été, moins coûteuses, mais de moindre qualité, et de rogner sur les coûts de distribution en abandonnant les États-Unis, la Scandinavie et l'Europe centrale, en gelant les passages en haute définition ou en TNT payante en Afrique, en supprimant la diffusion en onde moyenne vers le Moyen-Orient, sur la TNT outre-mer et, peut-être, en Île-de-France en 2020. Le groupe fonde quelques espoirs sur la participation de l'AFD pour de nouveaux programmes en langue africaine et de l'Union européenne pour des programmes numériques avec, mais ces développements ont un coût et cela ne répond que de façon adjacente au besoin de financement du socle des activités. Nous avions fondé des espoirs, l'année dernière, en imaginant rééquilibrer les allocations de la contribution à l'audiovisuel

Pourtant, nous continuerons à soutenir cette ambition parce que nous la croyons juste et parce que nous respectons les dirigeants et les personnels de ces médias, qui travaillent avec dévouement, talent et honnêteté, à promouvoir l'image et les valeurs de notre pays hors de ses frontières. Au-delà pèse évidemment une grande incertitude liée au projet de réforme de l'audiovisuel. Il est prévu dans le projet de loi de faire chapeauter France Télévisions, Radio France et France Médias Monde par une holding chargée de superviser et de coordonner les filiales, mais aussi de répartir le montant de la contribution à l'audiovisuel public qui lui sera désormais attribué, privant au passage le Parlement d'une partie du pouvoir de décision, que, mes chers collègues, nous exerçons ce soir même, ce qui n'est tout de même pas rien.

nous regrettons la baisse des moyens, lorsqu'elle a pour conséquence de remettre en question certaines missions de service public, qu'il s'agisse de l'existence d'une chaîne consacrée à la jeunesse, d'une autre tournée vers l'outre-mer, ou de l'arrêt de la diffusion de TV5 Monde dans les îles britanniques et en Europe et de France 24 en Amérique. En choisissant de manier de nouveau le rabot budgétaire sans discernement, le Gouvernement se prive d'une vision de long terme et contribue à la dégradation du climat social dans ces entreprises. Il n'est pas aisé, nous le savons, de faire évoluer le secteur des médias publics, surtout quand le ministère

Notre commission se mobilisera pour qu'une réforme du financement accompagne celle des structures. La holdingpublique France Médias Monde, née au Sénat, n'aura de sens que si une stratégie innovante peut s'appuyer sur des moyens identifiés et garantis dans le temps. Cette stratégie ne pourra se bâtir que sur la différenciation. C'est pourquoi je regrette que France Télévisions, Radio France et même France Médias Monde soient incitées par leurs tutelles à augmenter leurs ressources publicitaires pour boucler leur budget. moi, une décroissance de la publicité devra constituer une des clés du futur modèle économique de l'audiovisuel public. Le management par le stress budgétaire que vous avez mis en place, monsieur le ministre, aura eu pour mérite d'obliger France Télévisions et Radio France à engager véritablement la transformation de leur de leur modèle de production et à développer le numérique à tous les étages. L'enjeu pour les entreprises de l'audiovisuel public est, d'une part, de se conformer à la trajectoire budgétaire définie jusqu'en 2022, qui ne leur laisse que peu de marges de manoeuvre et, d'autre part, de participer à la définition des priorités stratégiques que France Médias sera chargée de mettre en oeuvre, souvent dans le cadre de partenariats avec d'autres acteurs. Ces entreprises et leurs salariés ont besoin de se mobiliser autour d'objectifs ambitieux : s'adresser à la jeunesse, défendre la francophonie, protéger la création et notre patrimoine audiovisuel et cinématographique. Le budget pour 2020 peut être considéré comme une potion amère, peu digeste ; je préfère l'envisager comme une diète salutaire, avant une remise à plat des missions, des outils et des moyens,

en chute libre, conséquence d'une transition numérique à laquelle les journaux n'ont, pour la plupart, pas su se préparer ; une crise morale, avec la remise en cause systématique, notamment sur les réseaux sociaux, d'une information traitée de manière professionnelle par des journalistes attachés aux faits.

des droits voisins, transposition de l'article 17 de la directive européenne. De cette réforme, le secteur de la presse attend légitimement beaucoup, mais l'attitude de Google est, pour l'instant, extrêmement frustrante ; elle appelle probablement une action européenne encore plus large. la modernisation de la distribution, sur laquelle, monsieur le ministre, vous avez apprécié, je crois, la contribution du Sénat à l'enrichissement d'un texte qui semble maintenant emporter l'adhésion du plus grand nombre.

Nous sommes très désireux de savoir où en sont les négociations avec vos homologues européens sur les droits voisins, et si une solution claire apparaît enfin

d'affirmer que la solidarité nationale ne s'exerce pas au bénéfice de la presse, même s'il pourrait être temps de réfléchir à une meilleure répartition des aides, pour mieux prendre le numérique. Je note, par ailleurs, des inquiétudes sur la question de la publicité ciblée, dont nous aurons à reparler dans le cadre de la discussion de la future loi audiovisuelle : vos annonces d'ouverture ont inquiété la presse régionale, mais sont jugées

d'un effet ciseaux mortifère, avec des dépenses en hausse et des revenus en baisse. L'impulsion donnée par le nouveau président de l'agence semble toutefois commencer à produire des résultats, comme en témoigne l'accompagnement de 17 millions d'euros que l'État a accepté d'accorder, dont 6 millions d'euros cette année.

animée (CNC) et 400 millions d'euros de crédits d'impôt, soit un montant total de près de 1,3 milliard d'euros. Je souligne avec force le caractère doublement stratégique de ce soutien public, à la fois pour des raisons économiques, au regard d'un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros,

Le nouveau président du CNC se trouve, pour sa première année, confronté à trois défis. Premièrement, la révision des dépenses pour améliorer l'efficacité de près de 150 dispositifs de soutien : le CNC doit dégager 25 millions d'euros d'économies, et l'épuisement de ses réserves laisse présager une baisse des investissements dans la production. la réforme de la fiscalité affectée, programmée l'année prochaine, mais dont l'article 62 du présent projet de loi de finances constitue la première étape. Troisièmement, la préparation de la future loi audiovisuelle, qui couvrira une myriade de sujets : relations avec les producteurs, obligations de financement des plateformes, diffusion des oeuvres à la télévision. Sur l'ensemble de ces sujets, nous resterons, monsieur le ministre, très mobilisés. J'ajoute que les menaces annuelles sur les crédits d'impôt « culture » n'aident pas à apporter de la sérénité au secteur. Sur ces questions, nous nous reverrons rapidement pour l'examen du projet de loi sur l'audiovisuel.

devrait enfin donner au neuvième art la place qu'il mérite, à la suite du rapport de Pierre Lungheretti. Nous en attendons beaucoup. Reste que la place singulière de la bande dessinée s'insère dans des conditions de travail et un régime social très tendus pour les auteurs. Si une solution a enfin été trouvée pour pérenniser la compensation de la CSG- je rappelle le combat mené conjointement par la présidente de notre commission, Catherine Morin-Desailly, et moi-même -, nous attendons avec impatience les conclusions du travail de M. Bruno Racine, en espérant que la spécificité du statut des auteurs soit enfin reconnue. Compte tenu de ces observations, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable sur les crédits du programme 334 de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». Mes chers

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le flot déversé à gros bouillons par les plateformes de l'internet, les réseaux dits sociaux et les chaînes d'information en continu a au moins pour avantage de susciter un intérêt croissant pour une information de qualité, des programmes qui parlent à notre intelligence, des confrontations d'idées et le respect du pluralisme de la pensée. Vous me permettrez d'interpréter de la sorte le succès historique du service public de l'audiovisuel, en remerciant les personnels qui l'ont bâti. Sans procéder à une revue de détail, je mentionnerai, pour l'exemple, les résultats exceptionnels de France Culture. Cette radio a porté, pour la première fois de son histoire, son audience à plus de 1,6 million d'auditeurs, soit une progression de 6 % en un an. Mieux encore, les téléchargements de ses émissions ont augmenté de 18 % en un an, ce qui représente un total de 31 millions d'écoutes à la demande ou une visite journalière pour 600 000 internautes. j'ai plaisir à souligner que l'émission est téléchargée plus de 3 millions de fois par mois ! Cette réussite sans précédent démontre que le pari de la qualité est toujours gagnant, et que les auditeurs apprécient des contenus exigeants. L'audiovisuel public contribue pleinement à sa mission de service public : apporter à nos concitoyens les informations, les idées et les connaissances dont ils ont besoin pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et ses évolutions fulgurantes. Nous cherchons, collectivement, à réduire dans notre société l'empire pernicieux des informations fausses, des préjugés menaçants et des théories complotistes. L'audiovisuel public est l'un des instruments de la riposte, car il a aussi pour mission d'instruire et d'éduquer. Enfin, je ne cache pas ma fierté devant l'intérêt que suscitent ces programmes à l'extérieur de nos frontières : ils contribuent ainsi au rayonnement de notre langue et de notre culture et apportent à celles et ceux qui subissent la propagande des gouvernements et des médias partisans les éléments d'une pensée critique et non asservie. Pour distinguer pareille réussite et encourager les personnels à poursuivre ce travail essentiel, nous eussions espéré que leur budget fût, à tout le moins, préservé. Il n'en est rien Ainsi, pour reprendre l'exemple de Radio France, sa dotation sera réduite de 5 millions d'euros l'année prochaine, alors même qu'elle doit financer sa conversion à la radiodiffusion numérique et poursuivre son programme de mise en ligne de ses contenus. On peut s'interroger sur l'objectif de ce nouveau plan de réduction d'emplois, quand on sait qu'un tiers des personnels de Radio France partiront à la retraite d'ici à 2025. Il est déraisonnable de penser que cette nouvelle saignée n'aura aucune conséquence sur l'offre de programmes ! Comment poursuivre l'engagement pour la qualité, après la suppression de seize postes de réalisateurs et de vingt postes de techniciens ? Les efforts consentis par les personnels de Radio France, considérables ces dernières années, ont permis à la structure de dégager un excédent d'exploitation l'an passé. La nouvelle purge obéit donc à d'autres finalités elle est à la fois une méthode de gestion sans ménagement et un moyen de réduire drastiquement et sur la longue durée les moyens publics consacrés à l'audiovisuel, quels que soient les succès d'audience, dont on nous avait pourtant dit qu'ils étaient les objectifs des précédentes réformes.

qu'un déficit hydrique de la vigne améliore la qualité du vin ; mais les salariés ne sont pas des plantes, et, à trop les pressurer, vous récolterez les raisins de la colère ! Du vinaigre ! Ils sont en grève aujourd'hui, et nous les soutenons. Dites plutôt la baisse d'un euro de la redevance audiovisuelle apparaît comme un moyen de pression supplémentaire. Elle intervient alors que le Gouvernement nous soumettra très prochainement un projet de loi d'ampleur, dont on nous explique qu'il sera pour l'État le moment d'une refondation des objectifs nationaux pour l'audiovisuel public. Le coup de rabot général que subissent tous les budgets pour l'année 2020 paraît d'autant plus violent et incompréhensible qu'il est aveugle et risque de fragiliser des entités déjà en grande difficulté- je pense en particulier à la composante internationale de l'audiovisuel public. la transformation de l'audiovisuel public que vous annoncez ne peut être définie ni conduite sans la participation effective des personnels. Elle doit être bâtie sur la confiance. Vous ne pourrez obtenir leur pleine mobilisation, si vous ne leur proposez pas un programme qui donne du sens à leur engagement pour leurs missions de service public. Au lieu de cela, votre budget pour 2020 leur révèle que la grande réforme à venir s'inscrira, dans tous les cas, dans un processus inflexible de contraction de toute la dépense publique, redevance comprise, et de réduction

Monsieur le président, monsieur le ministre,

et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création de l'art et de l'esprit qui l'enrichisse. La mission « Médias, livre et industries culturelles » du projet de loi de finances participe pleinement à la poursuite de cet objectif, à travers le soutien à la création musicale et littéraire et à la diffusion du savoir et des oeuvres par le biais des bibliothèques comme des médias. Le budget Le budget consacré à cette mission représente une enveloppe de 590,7 millions d'euros pour l'année prochaine, en augmentation de 2 % par rapport à la loi de finances pour 2019. Premier versant de cette mission, le programme 334, « Livre et industries culturelles », regroupe principalement les crédits destinés au financement de la politique du livre et de la musique enregistrée. Au premier rang des priorités de ce programme figure la politique de la lecture, premier moteur d'émancipation et de transmission entre les générations. l'année 2020 sera marquée par la consolidation du plan Bibliothèques mis en oeuvre par le Gouvernement selon les recommandations du rapport d'Erik Orsenna et Noël Corbin. Il s'agit de favoriser l'accessibilité de la lecture pour tous en accompagnant les collectivités territoriales dans leur effort d'extension des horaires d'ouverture et de création de nouveaux lieux de lecture, en particulier dans les zones quasi blanches, comme on en trouve encore en Dordogne, dans les Ardennes ou dans l'Aisne. de 16 500 lieux accueillant chaque année 27 millions de lecteurs, le réseau des bibliothèques est, avec celui de La Poste, le premier réseau public sur le territoire français. L'accès à la culture, au sens large, est la première vocation des bibliothèques et des structures dérivées comme les artothèques, qui offrent la possibilité d'emprunter des oeuvres d'arts visuels, et les Micro-folies, qui, à l'image du musée virtuel créé par Didier Fusillier, associent atelier numérique, espace scénique et conférences. La révolution numérique fait évoluer les usages au sein même de ces hauts lieux de diffusion du savoir, qui intègrent dorénavant postes informatiques, salles multimédias et médiathèques, autant de dispositifs contribuant à combler les fractures entre territoires et entre générations. Actuellement, 10 % seulement des bibliothèques desservant plus de 2 000 habitants proposent des postes informatiques adaptés aux personnes en situation de handicap. Nous devons poursuivre les efforts d'adaptation de ces lieux de lecture à tous les publics. L'année prochaine verra la création du Centre national de la musique, musique, doté d'un budget supplémentaire de 7,5 millions d'euros. Ces nouveaux moyens devraient permettre d'accompagner l'adaptation du secteur de la musique enregistrée à la transition numérique et à l'évolution rapide des modes de production, de distribution et de consommation. Deuxième versant de cette mission, le programme 180 regroupe les crédits consacrés au soutien de la presse et des médias. Le secteur, en cours de restructuration, bénéficiera l'année prochaine d'une augmentation de 1,6 % des crédits du programme, portés à 284,4 millions d'euros. Cette augmentation se concentre sur le soutien à l'Agence France Presse, troisième agence de presse à l'échelle mondiale et précieux rempart contre la désinformation relayée, entre autres, et massivement, par les réseaux sociaux. Le Gouvernement a fait le choix d'augmenter la subvention versée à l'agence de 6 millions d'euros pour financer son plan de transformation. Les crédits destinés au fonds d'aide au portage de la presse seront stabilisés, après une baisse de 5 millions d'euros l'année dernière, tout comme les crédits affectés au soutien des médias de proximité et des radios associatives locales. L'année 2020 marquera un tournant pour l'audiovisuel public, dans l'attente de la réforme présentée en conseil des ministres ce matin. matin. Elle sera également la deuxième année du plan d'économies appliqué au secteur, avec une baisse des crédits inscrits sur le compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » de 70 millions d'euros. L'essentiel de l'effort est demandé à France Télévisions et à Radio France ; il s'accompagne, pour les ménages, d'une diminution symbolique, de 1 euro, du montant de la contribution à l'audiovisuel public.

public. Ce matin, monsieur le ministre, vous avez présenté en conseil des ministres votre réforme, que vous nommez « projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère du numérique

qu'il ne peut y avoir de " souveraineté culturelle à l'ère du numérique " en baissant les moyens de l'audiovisuel public comme aujourd'hui, alors qu'il faut les augmenter ... » Nous sommes dans le sujet : 70 millions d'euros en moins

Dans ces conditions, à l'heure de la gigantesque révolution technologique mondiale, de la concurrence féroce des plateformes américaines sans foi ni loi et de l'intervention massive d'États comme la Chine et la Russie pour mettre en coupe réglée le marché de l'audiovisuel à l'échelle planétaire, comment voulez-vous assurer une quelconque souveraineté culturelle en baissant les moyens destinés à faire face ? Si, parfois, on peut faire bien avec peu de moyens, dans le domaine des médias à l'heure du numérique, pour l'instant, on ne peut pas, avec moins, faire qualitativement bien. Le non-sens est désolant : une baisse budgétaire préalable à l'élaboration d'une réforme qui a l'ambition de redessiner notre paysage audiovisuel. En d'autres on soumet l'ambition culturelle à un impératif budgétaire, au lieu d'inverser la démarche : soumettre la nécessité budgétaire à l'ambition culturelle et politique. À ce non-sens le Gouvernement en ajoute un autre, révoltant, en baissant de 1 euro la contribution citoyenne à l'audiovisuel. Ces 25 millions d'euros auraient pourtant été bienvenus pour alléger les contraintes de salariés méritants qui ont déjà consenti de grands efforts pour transformer leurs entreprises et mener un travail de qualité reconnu par les auditeurs, comme à Radio France. Je vous rappelle les faits : depuis 2012, France Télévisions a perdu 1 000

contesté par les grévistes prévoit 299 suppressions de plus d'ici à 2022. Pourquoi donc se priver de ces 25 millions d'euros ? Parce que, dites-vous, la redevance a rapporté plus, et que cet argent non prévu vient en surplus de la trajectoire budgétaire de baisse, arbitrairement décidée dans les bureaux de Bercy Quel dogmatisme ! Quel enfermement idéologique ! D'autant que, à l'heure où l'on ne cesse de nous montrer en exemple l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, pour nous vanter tantôt le sérieux de gestion, tantôt les bienfaits du libéralisme, et même le rayonnement de leur audiovisuel, avec notamment la BBC, il est bon de rappeler que notre redevance est déjà l'une des plus faibles d'Europe : nos voisins allemands paient 210 euros et les Britanniques 175 euros, là où vous ramenez la contribution française à 138 euros, après avoir bloqué l'année dernière son indexation sur l'augmentation du coût de la vie, pourtant acquise depuis 2010, quelles que soient les Je ne suis pas d'accord avec le rapport de mon collègue Leleux : ce ne sont pas les réductions budgétaires qui ont permis à l'audiovisuel public de se réformer, et les réductions de budget ne touchent pas uniquement les hauts salaires ; elles touchent, désormais, les programmes et les chaînes et entraînent une réduction de périmètre, avec la disparition de France qu'aucune politique de visibilité ne viendra compenser ! France 4 aussi est touchée, ce qui est destructeur pour le secteur de l'animation.

J'en veux pour preuve la suppression de postes de journalistes dans les territoires, alors même que l'actualité s'y déroule et que l'avenir réside dans l'ancrage territorial des médias ; alors même que BFM, qui recherche en général l'intérêt financier, ouvre antenne sur antenne au niveau local

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2019 s'achève sur un bilan riche et très positif. par l'adoption de plusieurs réformes majeures, comme celle du droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse, la réforme de la loi Bichet sur la distribution de la presse et la création du Centre national de la musique. Marc Twain, ce grand écrivain américain, se plaisait à dire que les actes en disent souvent plus long que les mots. C'est une réflexion qu'il est toujours bon, en particulier pour nous, parlementaires, de méditer. Chacun de vous connaît naturellement mon tempérament pondéré. Aussi, je n'aurai pas ici l'outrecuidance de comparer ce bilan législatif d'une année avec celui du quinquennat précédent. Pour en revenir aux actes, en particulier aux trois lois adoptées cette année dans le domaine des médias et des industries culturelles, je rappellerai deux faits. Le premier est que deux de ces trois textes ont été étudiés en première lecture au Sénat. C'est un fait suffisamment rare pour être souligné et consigné. Cela témoigne de la considération que vous portez, monsieur le ministre, à notre Haute Assemblée. Je me crois autorisé à vous en remercier en son nom. Le second fait, corollaire du premier, est que ces trois textes ont été

le Gouvernement a fait évoluer ces secteurs sans jamais se départir des valeurs qui président à la conduite du ministère de la culture depuis soixante ans : un secteur public fort, permettant de soutenir l'activité culturelle dans toute sa diversité et donnant un accès à la culture et à une information de qualité à tous nos concitoyens. Les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » et du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » pour 2020 sont guidés par ces mêmes objectifs. Certes, de réels efforts budgétaires sont demandés au secteur de l'audiovisuel public. Ce n'est pas une surprise : les objectifs de réduction ont été fixés il y a deux ans et étalés sur une durée de trois années. Des efforts de mutualisation ont notamment été demandés aux différentes sociétés de l'audiovisuel public, dans la perspective de rompre avec cette anomalie française qui veut que notre service public de l'audiovisuel soit représenté par pas moins de cinq sociétés, chacune ayant sa direction, ses fonctions support, et souvent, ses stratégies propres, pour ne pas dire personnelles, et ce à un moment où l'audiovisuel public doit faire face, non seulement à la concurrence de groupes français ou européens du privé toujours plus puissants, mais surtout, à deux grands opérateurs américains qui sont chaque jour plus présents sur le marché national. Je suis toutefois conscient des craintes actuelles des salariés de Radio France quant à l'avenir de leur emploi. Mais je suis aussi conscient que le numérique modifie profondément nos comportements, nos usages et nos liens sociaux, notamment en matière de communication. En un an, et en dépit des bonnes audiences de France Inter et de France Culture, le secteur radiophonique dans son ensemble a perdu plus d'un million d'auditeurs. Cette tendance ne peut aller qu'en s'accentuant. Face à ce changement, la seule réponse possible est de s'adapter aux nouveaux modes d'écoute, aux nouvelles attentes du public, tout en préservant sa spécificité. Les métiers de la radio, comme ceux de la télévision et du journalisme, sont en mutation profonde. L'audience tend de plus en plus à se fragmenter et à se délinéariser. Il y a une réalité assez cruelle, c'est que l'audience des médias tend à vieillir avec l'âge de ceux qui les font. La presse écrite, y compris la presse de qualité, a profondément renouvelé ses effectifs et ses modes de production au cours des dix dernières années, notamment pour s'adapter à la révolution numérique et à la transformation des usages.

public, comme certains ici le laissent entendre. Si tel était le cas, la très forte augmentation qu'a connue la CAP jusqu'en 2017 aurait dû conduire automatiquement à une consolidation des audiences et à un rajeunissement des publics des chaînes et des stations de l'audiovisuel public, ce qui n'a pas été le cas. Il ne s'agit pas de nier l'importance des questions budgétaires, même si, à première vue, face aux milliards déversés dans ce secteur par les grands opérateurs américains, les crédits de la mission et du compte spécial qui nous intéressent peuvent sembler modestes avec leurs 4,3 milliards d'euros pour 2020. Ces crédits visent d'abord à préserver le pluralisme des idées et la diversité culturelle dont se préoccupent peu les entreprises d'outre-Atlantique

désengagement de l'État à ce sujet, notamment si on observe les évolutions des dernières années dans ce domaine chez nos voisins européens. Dans une étude récente comparative présentée en février dernier, le Idate souligne en effet que les recettes annuelles des principaux groupes de l'audiovisuel public en Europe diminuent depuis 2012 en moyenne de 0,2 % par an. Un pourcentage moyen à mettre en parallèle avec les 0,18 % de baisse programmée en 2020 pour l'audiovisuel public français- année de plus forte réduction au sein de la trajectoire budgétaire qui avait été fixée pour trois ans. Nous sommes donc bien loin des coupes claires dénoncées par certains.

qu'il s'agit d'un chantier d'ampleur, car il s'agit ni plus ni moins que de remettre sur l'ouvrage une législation datant pour l'essentiel de 1986, et dont la refonte avait jusqu'à présent été abandonnée par nos prédécesseurs. Le groupe

pour l'excellence de son travail. Je concentrerai mon propos sur deux sujets : celui du modèle économique, et donc du financement de l'audiovisuel public, et celui, ô combien stratégique, de l'audiovisuel extérieur que l'on a parfois tendance à oublier en se concentrant sur les grandes masses budgétaires que représentent France Télévisions et Radio France. Le budget qui nous est aujourd'hui soumis est le dernier avant la grande réforme que nous attendons de longue date, réforme pour laquelle le Sénat a travaillé, considérant l'urgence d'adapter notre audiovisuel à la nouvelle donne numérique qui transforme les supports, les usages, les métiers, les organisations d'entreprise

notamment à l'amélioration de la gouvernance de l'audiovisuel public, via la constitution d'une holding visant à rapprocher, dans une vision stratégique, les quatre entreprises de l'audiovisuel public. Mais la gouvernance n'est pas tout. modèle économique de l'audiovisuel public reposant sur la modernisation de la CAP, élément essentiel d'une réforme qui ne peut être que systémique pour garantir la prévisibilité des ressources et l'indépendance d'un audiovisuel public libéré des dotations de l'État. Or, pour l'heure, sur ce chapitre, nous sommes dans l'incertitude, voire dans la confusion. En témoigne le sort réservé à la CAP. Le ministre de l'action et des comptes publics en a récemment proposé la suppression en même temps que celle de la taxe d'habitation (TH) à laquelle elle était adossée. Monsieur le ministre, vous vous étiez opposé à cette aussi, car nous considérons que l'audiovisuel public doit être principalement financé par une dotation publique pérenne et dynamique. Alors que nos voisins européens ont déjà modernisé leur redevance audiovisuelle, nous sommes depuis quelques années dans le yo-yo perpétuel, passant notre temps à la désindexer puis à la réindexer. Cette année, alors que la réforme de la TH n'est pas aboutie, on nous annonce une baisse de 1 euro de la CAP ! Si l'idée est d'alléger la fiscalité, en effet lourde pour nos concitoyens, attaquez-vous à l'impôt sur le revenu, pas à la CAP, d'autant que cette somme ne veut

désastreux quant à la légitimité de ce qui reste une contribution en échange d'un service identifiable, équivalente, somme toute, si elle était mensualisée, à un abonnement à une chaîne payante ou à une plateforme de Pour notre groupe, c'est l'incompréhension, d'autant que même sans cela, notre redevance reste la plus basse d'Europe. Oui, il faut faire aujourd'hui des gains de productivité-cela est demandé à tous-, mais il faut aussi avoir des marges de manoeuvre permettant de moderniser les entreprises,

déjà largement contribué à l'effort d'économies demandé. De ce fait, sa trajectoire est en décalage croissant avec les autres grands médias internationaux qui voient leur financement progresser. Je pense notamment à la, dont le directeur général a été auditionné par notre commission, mais aussi à d'autres médias proches de nos valeurs.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur l'audiovisuel public et les fonds qui lui sont consacrés. J'évoquerai d'abord le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique qui vient tout juste d'être présenté en conseil des ministres après de longs mois d'attente. En effet, si nous n'examinons pas aujourd'hui les crédits qui viendront en appui de cette réforme, on ne peut faire abstraction des enjeux qu'elle soulève. L'essor du numérique, de nouveaux usages, la véritable explosion d'offres venues bouleverser le paysage audiovisuel au niveau mondial nous obligent en effet à définir un nouveau cadre législatif et réglementaire.

Le Sénat a un rôle majeur à jouer dans cette réflexion. Certaines pistes avancées dans le rapport d'information de Jean-Pierre Leleux et André Gattolin en septembre 2015 ont d'ailleurs eu les faveurs du Gouvernement. Le projet de loi définit un modèle que notre rapport qualifiait de « BBC à la française permettant le regroupement des différentes sociétés de l'audiovisuel public et la mutualisation de leurs moyens. À la lecture des différents chapitres de ce projet de loi, si je retrouve les grandes lignes d'une organisation modernisée, je reste perplexe quant à l'ambition de ses Comme l'a souligné notre rapporteur pour avis Jean-Pierre Leleux, le problème semble être pris à l'envers : le Gouvernement définit une gouvernance, des rapprochements, des règles éparses concernant la publicité ou les rapports des acteurs en présence, mais sans déterminer au préalable ce que l'on attend du service public dans le nouveau paysage audiovisuel ce qui justifie son existence. Cette absence de réflexion sur les priorités est alarmante et augure mal des choix qui seront faits, notamment en matière de financement. Car enfin, si ces objectifs ne sont pas fixés, comment les moyens pourraient-ils être définis ? Le projet de loi reste muet, et vous également, monsieur le ministre, quant aux nouvelles sources de financement qui seront mises en place, celles-ci ne devant être définies qu'en 2021 et 2022. Ces derniers mois, la suppression de la redevance a été évoquée par le ministre des comptes publics, mais, à l'inverse, vous vous êtes prononcé par le passé pour un élargissement de son assiette. Le présent budget précède donc une reconfiguration qui demeure inconnue. Nous appelons de nos voeux de prochains éclaircissements. Pour en revenir aux crédits consacrés à l'audiovisuel public cette année, nous constatons une baisse de 69,2 millions d'euros, en cohérence avec la ligne définie et suivie par notre Haute Assemblée en 2018. En effet, une économie de 190 millions d'euros est demandée aux entreprises de l'audiovisuel public d'ici à 2022 au titre de la réduction des déficits publics, mais également afin de concentrer les moyens sur certains postes- je pense notamment au développement numérique. Cette stratégie d'austérité, qui succède à une forte augmentation des moyens de 2009 à 2017, a enclenché une réorganisation des services et la mise en oeuvre de diverses réformes. Certes, on peut s'interroger sur l'opportunité de maintenir cette trajectoire, alors que le fonctionnement de l'audiovisuel public, notamment de France Télévisions, sera prochainement revu par le Gouvernement. L'année dernière, la taxe Copé sur les télécoms a été définitivement affectée au budget de l'État au détriment de France Télévisions, alors qu'elle avait été créée pour compenser la suppression de de la publicité en soirée sur les chaînes de l'opérateur. Cette année, la contribution à l'audiovisuel public est diminuée de 1 euro, ce qui renforce l'impression de diète, même si la portée de cette décision est surtout symbolique. Je partage le sentiment de notre rapporteur Jean-Pierre Leleux, qui regrette cette baisse des moyens à la veille de la réforme annoncée, mais qui fait toutefois le choix difficile de ne pas s'y opposer. Les contraintes budgétaires ont en effet permis d'enclencher des mesures nécessaires de réorganisation et d'économie. Les entreprises de l'audiovisuel public ont incontestablement progressé dans la redéfinition de leurs priorités, ce qui n'aurait pas été possible si l'inflation de leurs moyens L'absence de réforme des sources de financement de l'audiovisuel public nous incite à poursuivre la même trajectoire. Pour ces raisons, notre groupe suivra l'avis de nos rapporteurs, et outre les crédits de la mission, adoptera ceux du compte spécial dédié à l'audiovisuel public. La parole

En particulier, grâce au Sénat, la France peut s'enorgueillir d'être le premier État membre à avoir transposé la directive européenne tendant à créer un droit voisin au droit d'auteur pour les agences de presse et les éditeurs de presse.

aisément à une grande pluralité de titres. Mes chers collègues, j'évoquerai tout d'abord les crédits attribués à l'audiovisuel public, plus particulièrement à France Télévisions. Notre rapporteur évoque à juste titre

de 70 millions d'euros l'an prochain, dont 40 millions pour France Télévisions -avant même de redéfinir les missions des structures visées, nous laisse assez dubitatifs. Nous continuons en outre de regretter les disparitions prochaines de France 4 dont l'offre jeunesse est précieuse, et de France Ô qui donne aux outre-mer une visibilité qu'il sera difficile de rétablir, alors que ces disparitions n'auront qu'une incidence mineure sur les comptes du groupe.

destinée à l'origine à compenser la suppression de la publicité en soirée sur France Télévisions, même s'il faut reconnaître que le parrainage remplace souvent la publicité Nous saluons enfin les excellents résultats de Radio France, et ce, en dépit des mesures d'économie, ainsi que l'accompagnement de l'État, à hauteur de 6 millions d'euros, apporté à l'Agence France Presse qui conduit actuellement une profonde restructuration. La situation de l'agence s'améliore lentement. Nous nous en félicitons. Ces outils nous sont précieux dans un contexte où la culture de l'immédiateté et la perte d'indépendance de certains médias desservent chaque jour davantage la qualité de l'information. Les industries culturelles continuent pour leur part de représenter un enjeu économique majeur en France. Livres, jeux vidéo, cinéma, musique : les productions françaises connaissent toujours un rayonnement international significatif, rendu possible par des politiques publiques spécifiques et un cadre protecteur où la régulation, à la demande des acteurs, est toujours forte. secteur de la culture demeurent stables : ils s'élèvent à 400 millions d'euros, dont 90 % seront absorbés par la production cinématographique et audiovisuelle. Après des années difficiles, le marché de la musique poursuit sa mutation et renoue avec la croissance grâce au. Certes, la rémunération des auteurs doit être adaptée à ce nouveau modèle économique. Le projet de loi sur l'audiovisuel nous permettra, je l'espère, de réduire l'écart aujourd'hui observé entre écoute et revenus. Le Centre national de la musique (CNM) offrira enfin à ce secteur, aujourd'hui encore largement éclaté, un nouvel outil pour faire face à des enjeux qui demeurent considérables. Tout comme vous, monsieur le ministre, nous sommes attachés à la réussite de ce projet qui vient enfin de se concrétiser. J'évoquerai pour conclure les aides de l'État à la presse. Ce secteur, qui doit faire face au défi de la numérisation, continue de voir chuter ses recettes de vente et ses recettes publicitaires. En dépit des réformes engagées, le secteur de la distribution demeure dans l'incertitude, avec un opérateur principal, Presstalis, dont l'avenir demeure très obscurci. Attachés à la proximité, les membres du RDSE se félicitent, dans un contexte morose, que la presse locale

Je ne m'étendrai pas longuement sur les crédits de la presse, le rapporteur pour avis Michel Laugier, dont je salue l'excellent travail, ayant déjà brossé un tableau d'ensemble du secteur. De ce panorama, nous voulons retenir les signaux positifs. Les grands opérateurs et les pouvoirs publics ont pris la mesure du choc numérique et ont commencé à s'y adapter. Ainsi avons-nous voté la loi relative à la modernisation de la distribution de la presse et la loi tendant à créer un droit voisin. Nous regrettons néanmoins qu'il n'ait pas été possible possible d'adosser Presstalis à un autre opérateur dans la loi. Je m'interroge également sur les conséquences en région de la contraction des aides versées à La Poste. Quant au droit voisin, la loi votée constitue un signal fort, mais compte tenu de la réaction de Google et de Facebook, l'offensive législative ne fait que marquer le début et industries culturelles » doivent donc être appréciés à l'aune des mutations structurelles en cours. Le soutien public à la presse demeure substantiel, et il ne faiblira globalement pas en 2020. Les aides directes sont concentrées sur la presse IPG, ce qui est une bonne chose, puisque ce secteur est celui qui a le plus souffert de la baisse des ventes et des recettes publicitaires. presse (Arcep) se déclare satisfaite du budget qui lui est alloué pour commencer à remplir sa nouvelle mission de régulation. Presstalis continue d'être soutenu à bout de bras par l'État, qui vient de débloquer un prêt de 90 millions d'euros. pour l'AFP, qui bénéficiera en 2020 d'une aide de 6 millions d'euros. Je dirai également un mot des crédits alloués aux industries culturelles. Comme le remarque très justement notre rapporteure pour avis Françoise Laborde, que je remercie également pour la qualité de son travail, le programme 334 qui les regroupe embrasse un champ particulièrement large, incluant le livre, la bande dessinée, la production audiovisuelle, dont le cinéma, la musique et le jeu vidéo. Les crédits du programme augmentent principalement du fait de la dotation d'amorçage du Centre national de la musique (CNM). La loi qui en porte création a été votée il y a déjà quelques mois, mais sa promulgation, intervenue le 30 octobre dernier, a été plutôt tardive. En effet, le CNM soulève toujours deux questions cruciales

dont le CNM aura besoin. Comment ce budget sera-t-il pérennisé ? Nous n'avons toujours pas d'assurance que les collectivités locales qui contribuent à l'animation et au financement de la politique musicale dans les territoires ne soient pas les grandes oubliées dans la gouvernance du CNM.

l'inéluctabilité de la baisse des dépenses du CNC conduit à penser que nous arrivons au bout d'un cycle : il faudra trouver un autre modèle de financement

va être vital pour le monde de la culture dans les années à venir, ce qui incite à ne surtout pas en réduire la voilure fiscale, comme le fait malheureusement le présent projet de loi En conclusion, malgré les incertitudes qui pèsent tant sur le secteur des médias que sur celui des industries culturelles, le groupe Union Centriste votera le présent budget, qui a au moins le mérite d'en accompagner les mutations.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans son discours du 20 mars 2018, le Président de la République avait fait part de son ambition pour la francophonie. Quelques mois plus tard, l'audiovisuel extérieur de la France, vecteur de la francophonie et outil indispensable au rayonnement de notre pays, était considérablement affaibli dans le projet de loi de finances pour 2019. France Médias Monde, opérateur majeur qui atteint chaque semaine près de 130 millions d'auditeurs et de téléspectateurs, subissait une baisse de crédits de 1,6 million d'euros. Cette année, la dotation allouée est encore en baisse de 1 million d'euros. Alors que France Médias Monde a déjà réalisé des efforts importants en matière de réduction de coûts- loyer, salaires -, ainsi que dans la recherche de nouveaux financements- Agence française -tentant de compenser la baisse de la redevance, le Gouvernement souhaite que soit menée une réflexion stratégique pour « garantir les meilleures conditions d'accomplissement de ses missions prioritaires ». Il s'agit donc de faire plus avec toujours moins de moyens, comme à Radio France, comme à l'hôpital et comme dans de nombreux services publics. Malheureusement, le résultat de cette politique est connu et inévitable : une baisse de la qualité des services. L'affaiblissement de France Médias Monde est d'autant plus inquiétant que de nombreux pays renforcent considérablement leur audiovisuel extérieur. Ainsi, la BBC bénéficie d'un budget de 436 millions d'euros

Ils souffrent tous d'une sous-dotation, de même que TV5 Monde, qui a subi une baisse de 1,2 million d'euros l'année dernière, baisse qui n'est pas compensée cette année. Je ne peux que regretter ces incohérences et la dichotomie entre les discours et la réalité des moyens alloués. Des efforts considérables sont déployés par les équipes de l'audiovisuel extérieur pour développer de nouveaux projets. Pour autant, la dégradation de leurs moyens entache fortement leurs conditions de travail. Je pense notamment à la question délicate de la protection sociale des journalistes pigistes à l'étranger qui n'est, à ce jour, pas encore réglée, monsieur le ministre. Les journalistes travaillant hors de France sont pourtant eux aussi les garants d'une information libre, pluraliste, et d'une certaine idée de la démocratie. En conclusion, la trajectoire budgétaire de l'audiovisuel extérieur n'est pas à la hauteur des ambitions de notre pays.

notre rapport à l'information, à la presse, aux médias et nos pratiques culturelles sont aujourd'hui bouleversés par la révolution numérique ; par la démultiplication des acteurs, des écrans, des formats, des contenus ; par la diversification des moyens de les lire, de les écouter, de les visionner. En même temps qu'il fait émerger des opportunités nouvelles, le numérique remet en cause des pans entiers de l'économie de la culture et des médias. Notre responsabilité est de faire du numérique une chance, et non une menace ; de le rendre synonyme d'enrichissement, et non d'appauvrissement ; de de faire en sorte que notre culture soit consolidée, et non précarisée. C'est en ayant en tête cette idée, cet objectif, cette obsession, que nous avons conçu le budget du ministère de la culture pour l'année 2020. Sur les 60 millions d'euros de crédits budgétaires supplémentaires dont bénéficiera le ministère, 9 millions d'euros iront à la mission « Médias, livre et industries culturelles

Nous poursuivrons notre action en faveur du développement de la lecture, laquelle ne doit pas être cantonnée au seul cadre scolaire. À l'heure de la diversification des sources d'information et de la prolifération des « infox », il ne faut plus seulement apprendre à lire, il nous faut aussi éduquer à l'image. est l'objectif du plan d'éducation aux médias et à l'information, dans lequel l'audiovisuel public s'engagera afin de lutter contre les infox, grâce, entre autres, à la plateforme de décryptage « vrai ou ».

Nous soutiendrons son plan de transformation, à hauteur de 4,5 millions d'euros supplémentaires en 2020. C'est un effort considérable. Nous accompagnerons également les missions d'intérêt général de l'AFP, en revalorisant leur financement à hauteur de 1,5 million d'euros. Cette information fiable, pluraliste, de qualité, nous n'aurons de cesse de la soutenir. Nous n'aurons de cesse de défendre la presse, son indépendance, sa liberté, parce que sans elle, il n'y a pas de démocratie. Les aides à la presse seront confortées en 2020. Avec mes homologues européens, je mène un combat pour faire respecter le droit voisin.

doit rester en première ligne sur ce sujet. Derrière le droit voisin, c'est l'avenir du journalisme qui se joue ; c'est la préservation des moyens des éditeurs et des agences de presse ; c'est la protection de leur indépendance, de leur capacité d'informer, tout simplement, d'une façon professionnelle. Aujourd'hui, la valeur créée est captée par les géants du numérique : c'est inacceptable, et il faut remédier à ce problème. Vous savez que l'Autorité de la concurrence a été saisie par les éditeurs de presse et qu'elle

est notamment l'enjeu de la révision de la loi Bichet. À cet égard, je remercie Michel Laugier de son travail, ainsi que tous les parlementaires qui se sont mobilisés pour cette réforme.

l'État est pleinement mobilisé, comme il l'a été dans le passé, pour assurer la pérennité du système de distribution de la presse. L'Arcep, qui, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi Bichet, est compétente pour la régulation du secteur, est également pleinement mobilisée. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de la suite du travail que nous effectuons avec la totalité de la filière, dans le cadre du plan de filière sur lequel Bruno Le Maire Renforcer la cohésion des territoires, c'est aussi moderniser nos services publics culturels de proximité. Telle est l'ambition que nous portons avec le plan Bibliothèques, dont le budget augmentera l'année prochaine. Le bilan qui est en train d'être réalisé est tout à fait

Cela implique d'accompagner la structuration des industries culturelles et créatives, notamment. Tel est le sens des états généraux des industries culturelles et créatives lancés la semaine dernière avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

recevra 7,5 millions d'euros dès 2020, son budget ayant vocation à monter en puissance pour atteindre 20 millions d'euros par an en régime de croisière. Par ailleurs, 2020 sera l'année de la bande dessinée, certains d'entre vous

ambitions : une ambition de dynamisme et de souveraineté culturels, afin de permettre le développement de la diversité, de la créativité, ainsi que le rayonnement de l'audiovisuel et du cinéma français

de loi établira un cadre adapté à la télévision, à la radio et à l'audiovisuel du XXI siècle, en tenant compte de la révolution numérique. Je rappelle que la loi de 1986 a été pensée et votée avant l'ère d'internet.

Il n'est pas question de leur tourner le dos ou de s'opposer à elles. Ce projet de loi se fera non pas contre les plateformes, mais avec elles. Nous devons assurer l'équité entre les différents acteurs, rééquilibrer les règles du jeu, entre les chaînes de télévision et les nouveaux services. C'est un combat qui exige détermination et persévérance, et qui nécessite des moyens- nous aurons l'occasion bien sûr de reparler du financement de l'audiovisuel public. Nous pouvons

Amazon, je le rappelle, détruit chaque année 20 000 emplois de plus qu'il n'en crée, quand les petites librairies de quartier, elles, ont perdu 1 500 emplois, soit une baisse de 12 %.